La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 4 juin 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger les victimes de violences conjugales n° 483, rapport n° 482). Notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle que tous les orateurs, y compris les membres du Gouvernement, s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune.

j'ai pu adresser aux procureurs généraux par circulaire une instruction leur demandant de déployer l'ensemble de notre arsenal répressif afin de faire preuve de la plus grande fermeté à l'égard des auteurs de ces violences, mais aussi afin de mieux protéger les victimes, par exemple en utilisant largement les téléphones grave danger. De 300 appareils distribués en février 2019, nous sommes ainsi passés à plus de 1 000 aujourd'hui. Cette volonté, portée par l'ensemble du Gouvernement, s'est exprimée tout au long de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Au-delà des dispositifs de signalement spécifiquement organisés par mes collègues ou de la création d'une plateforme d'hébergement et de suivi des conjoints violents, j'ai pu prendre diverses mesures. J'ai ainsi tenu à ce que les violences conjugales demeurent un contentieux prioritaire effectivement traité par les juridictions pendant la période de confinement. L'ordonnance de protection a donc figuré parmi les procédures d'urgence inscrites dans les plans de continuation d'activité des tribunaux avec, selon un schéma de procédure fixé par circulaire, un traitement des nouvelles demandes dans un délai de six jours, conformément à la loi du 28 décembre 2019. J'ai par ailleurs veillé à faciliter les démarches des victimes de violences conjugales en prolongeant toutes les ordonnances de protection dont le terme était prévu entre le 12 mars et la et la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce augmenté d'un mois afin de tenir compte du ralentissement de l'activité des juridictions. Ainsi, la loi du 11 mai 2020 ayant prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, une ordonnance de protection qui, par exemple, devait s'achever le 1 avril 2020 continuera à s'appliquer jusqu'au 10 octobre 2020. Je connais aussi, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l'engagement qui est le vôtre dans cette lutte contre les violences commises au sein du couple. Ces enjeux concernent

Ce texte marque un pas important dans ce combat, car il renforce les moyens de lutte contre ces violences en améliorant le traitement des requêtes en ordonnance de protection, en favorisant l'aménagement de l'autorité parentale en présence d'un crime conjugal, notamment en instituant la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale d'un parent poursuivi ou condamné pour crime commis sur la personne de l'autre parent, en permettant également le déploiement du bracelet anti-rapprochement et en étendant le champ d'application du téléphone grave danger. J'ai tenu à présenter l'ensemble de ces dispositions, pour la plupart d'application immédiate, dans une circulaire datée du 28 janvier 2020 adressée Cette circulaire comporte des instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales, impulsé et piloté par ma collègue Marlène Schiappa. mesures sont relatives à l'accompagnement des victimes, au suivi des auteurs et à l'organisation des juridictions en faveur d'une filière d'urgence dédiée au traitement des violences conjugales. La loi de décembre 2019 met spécifiquement l'accent sur les ordonnances de protection et sur les nouvelles mesures qui peuvent être prononcées dans ce cadre. On peut citer : l'interdiction de se rendre dans certains lieux où se trouve de façon habituelle la victime ; la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur ; et la possibilité pour celui-ci de suivre le stage de responsabilisation pour la pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Ces nouvelles mesures ont été favorablement accueillies dans les juridictions qui se mobilisent pour construire, sur ce sujet, des projets de juridiction. Les services du ministère de la justice se sont également mobilisés pour formaliser la nouvelle procédure de délivrance des ordonnances de protection afin de permettre aux juridictions de statuer dans le délai de six jours souhaité par le législateur. Le décret portant application des articles 2 et 4 de la loi du 28 décembre 2019 a ainsi été publié le 28 mai dernier. Ce décret supprime la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, qui manifestement était devenue incompatible avec le délai de six jours. Il unifie également les modalités de saisine du juge au profit de la requête signifiée. Le décret précise les conditions procédurales nécessaires au respect du délai de six jours tout en garantissant une procédure contradictoire, fondement de notre procédure civile. Je sais que d'aucuns trouvent ces procédures trop strictes, mais c'est un décret qui tend à garantir la mise en oeuvre des engagements du Gouvernement et la volonté du législateur. Des échanges sont en cours afin de faciliter l'accès aux huissiers pour assurer leur signification dans les délais requis. Mes services travaillent en outre à un possible doublement du délai de signification. Dès demain, une rencontre avec des professionnels va nous permettre d'avancer positivement sur ce sujet. Le décret crée, par ailleurs, une passerelle entre la procédure d'urgence de l'ordonnance de protection et la procédure au fond, relative à l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Grâce à cette passerelle, le demandeur n'aura pas à former une nouvelle demande en justice en cas de rejet de sa demande d'ordonnance de protection et il pourra obtenir rapidement une décision au fond. Toujours trop peu délivrée, même si le nombre est en augmentation constante, j'ai souhaité constituer un comité de suivi de l'ordonnance de protection dont j'ai confié la présidence à Ernestine Ronai. Ce comité pourra nous aiguiller sur les améliorations toujours possibles de nos pratiques. Notre engagement collectif va encore plus loin. De nombreuses propositions issues du Grenelle contre les violences conjugales, organisé par le Gouvernement, ont été formulées. Elles sont toutes destinées à mieux prévenir et à mieux réprimer ces violences. Certaines exigent des modifications de nature législative, qui trouvent leur expression dans la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales que nous allons examiner aujourd'hui. Nourries des réflexions et des concertations menées au sein des groupes de travail mis en place par Marlène Schiappa dans le cadre du Grenelle, ces propositions intègrent le cadre du Grenelle, ces propositions intègrent des notions indispensables à la bonne compréhension et au traitement adapté de ces violences indignes de notre civilisation. Ainsi, le phénomène d'emprise, ce mécanisme qui place la victime sous la domination et la dépendance de son conjoint, est particulièrement pris en compte. Il permet de comprendre le silence des victimes et leur comportement craintif, qui fait croire à tort à une acceptation de leur sort. C'est pourtant cette emprise qui les cloue cloue auprès de leur bourreau et peut les entraîner vers la mort. La proposition de loi que vous examinez aujourd'hui modifie le code civil, le code pénal et le code de procédure pénale en complétant la loi du 28 décembre 2019 sur des points importants, en vue de renforcer davantage encore la protection effective des victimes de violences familiales, qu'il s'agisse des parents ou des enfants. Sur le plan pénal, tout d'abord, la proposition de loi se concentre sur trois axes majeurs. premier axe est de faciliter le signalement des violences conjugales. À cette fin, dans les cas de violences d'une particulière gravité et qui démontrent la situation d'emprise de la victime, la proposition de loi donne la possibilité aux médecins ou aux autres professionnels de santé de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République, même s'ils n'ont pas réussi à obtenir l'accord de la victime. Je me réjouis que ces dispositions importantes aient reçu l'accord de votre rapporteur et de votre commission des lois, qui les ont non seulement approuvées, mais également améliorées. Les modifications apportées au texte, sur l'initiative de votre rapporteur dont je souligne ici la qualité du travail, mettent en effet très utilement en évidence le fait que le médecin appréciera en conscience s'il doit ou non procéder à un signalement. Ces modifications clarifient également la notion d'emprise pour que le médecin puisse plus aisément apprécier si un signalement est ou non justifié. Le deuxième axe est d'améliorer les procédures pénales concernant ces infractions. Dans ce cadre, est prévue l'interdiction absolue du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales, ce qui répond à une demande ancienne et répétée des associations et se justifie par la situation d'emprise dans laquelle se trouvent le plus souvent les victimes. L'efficacité de la procédure est par ailleurs accrue en permettant au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner, en cas de violences conjugales, dans le cadre d'un contrôle judiciaire- et donc avant toute condamnation -, la suspension du droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants, y compris en l'absence de violences directes à leur encontre. Dans le même esprit est renforcée la possibilité pour les enquêteurs de saisir des armes, notamment au cours d'une procédure pour violences au sein du couple, afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées par la personne mise en cause. Le troisième axe, toujours sur le plan pénal, vise à améliorer les incriminations et à renforcer la répression. Cela se traduit notamment par les points suivants. sera réprimé de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le harcèlement au sein du couple qui aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire. Ensuite, les comportements d'espionnage au sein du couple seront plus largement incriminés. la lutte contre l'exposition de mineurs à la pornographie, notamment sur des sites internet, sera améliorée par la précision apportée à l'article 227-24 du code pénal selon laquelle le délit sera constitué, y compris si l'accès d'un mineur à des messages pornographiques résulte d'une simple déclaration de de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins 18 ans. Enfin, le fait de donner mandat à une personne de commettre des crimes tels que le viol ou le délit d'agression sexuelle sur un mineur sera puni à titre autonome, y compris si le crime ou le délit n'a été ni commis ni tenté. Cela permettra notamment de poursuivre et de condamner des personnes qui visionnent sur internet des sévices sexuels qu'ils ont commandités et qui sont commis sur des mineurs à l'étranger. mineurs à l'étranger. Sur le plan civil, la proposition de loi prend en compte les conséquences dévastatrices des violences commises au sein du couple à l'égard de la victime, mais aussi de la famille. Deux propositions sont faites en ce sens. Concernant l'obligation alimentaire tout d'abord, en cas de violences conjugales graves, le texte exclut toute possibilité de voir les enfants, victimes indirectes, contraints à soutenir financièrement celui qui a été condamné. Comme le propose la commission des lois du Sénat, ce sont l'ensemble des obligés alimentaires qu'il convient de protéger en cas de crime au sein de la famille. Viennent ensuite des propositions concernant l'indignité successorale la lutte contre les violences au sein du couple, voire plus largement au sein de la famille, se poursuit sur le plan successoral. La proposition de loi engage une réflexion sur l'indignité successorale : le conjoint n'est plus légitime à hériter lorsqu'il a commis des violences graves envers le défunt. Ainsi que vous l'avez également décidé, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, dans la loi du 28 décembre 2019, le port du bracelet anti-rapprochement, dispositif qui sera déployé à partir de septembre 2020, pourra être non seulement ordonné par un juge pénal, mais aussi prévu par un juge civil. À cet égard, je soutiens l'amendement défendu par le groupe LaREM, tendant à assurer un suivi efficace de la personne à protéger lorsque le porteur du bracelet s'approche ou se maintient dans la zone dangereuse, en violation de la décision civile d'ordonnance de protection. Je me félicite de nouveau du travail effectué par votre commission, qui a accepté les dispositions proposées en les complétant souvent utilement sur un certain nombre de points. Je partage également votre remarque sur l'organisation des débats. J'aurais moi aussi préféré un texte unique, mais la proposition du député Aurélien Pradié est arrivée avant la fin du Grenelle, à un moment où de nombreux points faisaient encore l'objet de concertations. Parce que ce texte permettait la mise en oeuvre rapide de propositions qui faisaient déjà l'objet d'un consensus, le Gouvernement et la majorité l'ont pleinement soutenu. Tout ce qui peut contribuer, en effet, à lutter contre les violences intrafamiliales que nous combattons en commun ne peut être que positif. Grâce à votre engagement et au travail du Gouvernement, de premiers résultats se dessinent. Le nombre de demandes d'ordonnance de protection est passé de 3 300 en 2018 à 3 930 en 2019, soit une augmentation de plus de 21 %. Elle paraît encore plus importante si l'on note qu'il n'y en avait que 2 975 en 2016. Il reste cependant beaucoup à faire ! Plus significatif encore probablement, même s'il convient d'être extrêmement prudent, on déplore à ce stade 36 homicides conjugaux en 2020, contre 150 sur l'ensemble de l'année 2019. Ce n'est évidemment pas une victoire, et nous ne saurions en aucun cas nous satisfaire de ces chiffres toujours glaçants, mais cette diminution du nombre de faits constatés est sans doute un marqueur de la pertinence des dispositifs qui ne sont pas encore totalement déployés, mais que nous avons construits ensemble et mis en oeuvre. Ces éléments, je le crois, donnent de l'espoir et renforcent notre volonté. C'est bien en ce sens qu'il faut continuer à travailler ensemble, et je vous en remercie

des professionnels, des associations, des familles se mobilisent de longue date contre les violences conjugales. Heureusement, depuis quelques années, on observe que cette mobilisation va au-delà des sphères militantes qui, habituellement, luttent contre les violences conjugales. La société se réveille enfin- médias, politiques, citoyens -et finit par rejeter massivement ces faits que l'on appelle désormais par leur nom : les féminicides. C'est la raison pour laquelle, dès 2017, le Président de la République a décidé de faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat et d'agir sur ces questions. Les associations de longue date étaient mobilisées pour demander au Gouvernement d'organiser un Grenelle des violences conjugales. Le Gouvernement a considéré qu'il était temps de rassembler les personnes qui travaillaient jusque-là parfois séparément dans la lutte contre les violences conjugales : les personnels soignants, la police, la gendarmerie, le monde de la justice, les associations, les familles de victimes. Plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs participé à ce Grenelle des violences conjugales et se sont réunis à Matignon le 3/9/19, date choisie en référence à la ligne d'écoute du 3919 pour mieux la faire connaître. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a alors lancé un travail inédit à Matignon composé de onze groupes pour formuler des propositions sur des thématiques aussi variées que les violences intrafamiliales, l'éducation, la santé, la sphère professionnelle, les outre-mer, le handicap, l'accueil en commissariat et en gendarmerie, l'hébergement, la justice, les violences psychologiques, l'emprise et, enfin, les violences économiques. Pendant trois mois, ces groupes de travail se sont réunis et ont avancé ensemble afin de trouver des solutions pour mieux protéger les femmes face aux violences conjugales, pour mieux prévenir ces violences conjugales, mieux sanctionner leurs auteurs et pour éviter que nous continuions simplement à battre le décompte des féminicides. Connu par 9 % seulement de la population avant le Grenelle des violences conjugales, grâce à la mobilisation collective, le numéro du 3919 est désormais connu par plus de 65 % de la population. Le 25 novembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé les mesures retenues par le Gouvernement dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. L'ensemble des propositions restituées fin octobre par les responsables des groupes ont été alors reprises par le Gouvernement. Ce Grenelle des violences conjugales a donné lieu à plus d'une cinquantaine de mesures de politiques publiques. Certaines ne relèvent pas de la loi directement ; d'autres, oui. Elles sont devenues ou deviendront réalité grâce aux deux propositions de loi évoquée à l'instant par Nicole Belloubet. La première proposition de loi, vous la connaissez, vous en avez débattu, c'est celle qui a été adoptée sur l'initiative du député Les Républicains Aurélien Pradié.

Comme nous le disions précédemment, cette mobilisation collective de la société civile, des experts, des préfets, des élus a permis de travailler à des mesures concrètes, dont certaines ont pris effet immédiatement pour agir contre les violences conjugales. Par exemple, avec Ernestine Ronai et les associations, nous avons mis en place une grille d'évaluation du danger que nous avons présentée avec le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner. Cette grille s'accompagne d'une nouvelle formation, d'une durée de 120 heures en formation initiale, pour les policiers et pour les gendarmes, afin que les femmes soient mieux accueillies encore dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie.

prévues dans cette proposition de loi, ils pourront désormais mieux signaler les violences conjugales subies par les victimes et peut-être parfois même leur sauver la vie. On entend souvent dire qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les trois jours. En réalité, lorsqu'on étudie sérieusement les chiffres et les dossiers, on s'aperçoit que le premier mode opératoire pour les féminicides en France est l'arme à feu. C'est pourquoi il nous a semblé important de saisir ces armes. Cela n'évitera pas tous les féminicides, mais cela pourra sans doute en empêcher. Grâce à cette action Grâce à cette action du Grenelle des violences conjugales, grâce à ces nouvelles dispositions législatives, les policiers, les gendarmes pourront désormais saisir les armes des auteurs de violences dès le dépôt de plainte pour empêcher les féminicides. Comme l'a rappelé la garde des sceaux, Nicole Belloubet, dont je voudrais ici saluer l'engagement total contre les violences conjugales et pour protéger les femmes, nous aurons à déployer le nouveau dispositif des filières de l'urgence, afin que les affaires de violences conjugales soient traitées plus rapidement et plus efficacement. Enfin, la société tout entière commence véritablement à prendre en compte la situation des enfants dans les cas de violences conjugales. Avec le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, qui nous rejoindra, nous portons des mesures de protection des enfants, notamment celles qui prévoient d'aménager l'exercice de l'autorité parentale. Je sais à quel point ces mesures vous tiennent à coeur, madame la rapporteure. Ce texte vise également à prévoir de décharger les descendants de leur obligation alimentaire envers le parent condamné, comme cela est demandé d'ailleurs depuis des années par différentes associations. Le terreau des violences conjugales est un phénomène de domination d'un membre du couple sur l'autre. Pour la première fois, il vous est proposé de faire entrer la notion d'emprise dans la loi. Je voudrais donc ici saluer saluer notamment le travail et l'engagement de l'ex-avocate Yael Mellul, qui a piloté ce groupe de travail et qui a oeuvré pour faire en sorte que ce que l'on appelle le « suicide forcé » soit reconnu désormais comme une circonstance aggravante. Quand nous avons lancé le Grenelle des violences conjugales, certaines voix se sont élevées pour souligner que l'État n'avait pas encore engagé une vraie politique de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Avec la garde des sceaux, nous avons écouté ces voix et nous avons décidé de travailler sur cette question : nous avons donc décidé d'ouvrir d'ici à la fin du quinquennat deux centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales par région. Nous avons d'ores et déjà lancé un appel à projets et plusieurs territoires y ont répondu. Nous souhaitons que, dans chaque territoire, on puisse prendre en charge les auteurs de violences conjugales, comme cela se pratique déjà à Arras. Prendre en charge les auteurs, c'est diminuer la récidive et, donc, c'est protéger les femmes face aux violences conjugales.

s'apercevant qu'ils ne peuvent pas gérer leurs accès de colère et de violence puissent être écoutés, puissent être pris en charge et puissent bénéficier d'un accompagnement psychologique. Je vous l'annonce aujourd'hui, cette ligne d'écoute est en train de passer la barre des 500 appels depuis sa mise en oeuvre le 6 avril Avec la garde des sceaux, nous l'affirmons, l'éviction du conjoint violent est une mesure fondamentale. Grâce à la mise en oeuvre d'une plateforme d'hébergement spécifique avec le Groupe SOS, en liaison avec les parquets, les conjoints sont désormais éloignés en moins de trois heures, contre quarante-huit heures auparavant. Une centaine d'auteurs ont d'ores et déjà, depuis le début du confinement, été écartés du domicile grâce à cette mobilisation et à ce partenariat. Notre priorité est de mettre fin à la cohabitation entre l'agresseur et la victime. Il importe de sortir l'homme violent du foyer ou de mettre à l'abri toutes les femmes qui en ont besoin.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ces quelques mesures phares du Grenelle des violences conjugales sont complétées par des dizaines d'autres qui font l'objet d'un suivi rigoureux et régulier dans leur application et dans leur déploiement. C'est à cet effet, ce matin, que j'ai réuni à Matignon les pilotes des onze groupes de travail du Grenelle des violences conjugales, qui poursuivent leurs efforts. Je tiens à les en remercier et à saluer le travail entrepris par l'ensemble des administrations dans la bonne réalisation des mesures, en coordination avec l'ensemble des ministères concernés et le service des droits des femmes et de l'égalité. Grâce à leur implication, un tiers des mesures du Grenelle des violences conjugales est d'ores et déjà réalisé. Un autre tiers est en cours de déploiement. Le dernier tiers poursuit sa préparation, notamment en ce moment même, ici, avec vous, avant de pouvoir être déployé. Le confinement a été une épreuve collective qui est venue percuter l'histoire personnelle et familiale de chacun. Vous le savez, il y a eu cinq fois plus de signalements de violences conjugales sur le portail « arretonslesviolences.gouv.fr » et 36 % de signalements en plus auprès des forces de l'ordre. Nous nous sommes mobilisés et la magistrate Élisabeth Moiron-Braud me remettra en juillet les résultats de sa mission sur l'évaluation de la prévalence des violences conjugales pendant le confinement. Nous notons d'ores et déjà que, s'il y a eu davantage de signalements, il y aurait eu- je parle au conditionnel et avec prudence -moins de féminicides qu'habituellement. Je voudrais également ici remercier les partenaires privés de leur engagement auprès des associations, puisque des partenariats nous ont permis d'ouvrir 90 points d'écoute et d'orientation avec les associations pour les femmes victimes de violences conjugales. Je pense, notamment, au centre d'entraînement du club de football de l'OM, qui a été un exemple d'engagement pendant le confinement puisqu'il a mis ses locaux et une partie de son personnel à disposition pour loger les femmes victimes de violences conjugales, en partenariat avec les services de l'État. Vous le savez, le signalement par SMS au 114 a été rendu possible et nous avons créé un fonds d'urgence de 1 million d'euros afin de soutenir davantage les associations et financer 20 000 nuitées pour les victimes de violences conjugales. Pour finir, je salue ici l'engagement des parlementaires de tous les bords pour mener à bien ces travaux lors de la tenue du Grenelle des violences conjugales. Vous êtes nombreuses et nombreux sur ces travées à avoir participé aux quelque 180 événements locaux qui se sont tenus partout en France et qui ont réuni plus de 4 500 personnes. Je voudrais particulièrement remercier les sénatrices et les sénateurs de la commission des lois, notamment Mme la rapporteure, Marie Mercier, ainsi que les sénatrices et les sénateurs de la délégation aux droits des femmes du Sénat pour les enrichissements qu'ils ont pu apporter au texte.

collègues, encore, me direz-vous, une loi sur les violences conjugales ! Et toujours tant de violences : 36 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Aussi, quelques mois seulement après la promulgation de la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, portée par le député Aurélien Pradié, le Sénat est saisi d'une proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, présentée par deux députés de la majorité, Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha. Ce nouveau texte a pour ambition d'inscrire dans la loi certaines préconisations du Grenelle contre les violences conjugales, dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 novembre dernier. Il comporte aussi des mesures visant à protéger les mineurs ou à prévenir les violences en général. Sur le plan de la méthode, la commission regrette que deux textes se soient ainsi succédé à quelques mois d'intervalle. L'examen d'un texte unique, déposé après le Grenelle, nous aurait permis d'avoir un débat plus cohérent, avec une vision globale de la politique de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Le calendrier qui nous a été imposé n'a pas non plus facilité notre travail : nous avons été informés il y a tout juste deux semaines que ce texte serait examiné aujourd'hui en séance publique, ce qui nous a laissé peu de temps pour achever notre cycle d'auditions, suspendu pendant la période du confinement.

Je sais que la délégation sénatoriale aux droits des femmes, dont je salue la présidente, a cependant mené un travail de veille sur le sujet au cours des trois derniers mois, ce qui nous permettra de disposer bientôt de premiers éléments d'information très pertinents. Sur le fond, la commission accueille favorablement la plupart des mesures qui figurent dans cette proposition de loi. Il nous semble toutefois que l'on approche un peu les limites de ce qu'il est possible de faire en matière législative, l'arsenal juridique étant déjà très étoffé. Beaucoup de dispositions du texte consistent en des ajustements, des clarifications, des précisions, que nous n'avons pas de raison de rejeter mais qui ne nous semblent pas non plus de nature à renforcer de manière significative la lutte contre les violences conjugales. Le texte propose, tout d'abord, d'interdire le recours à la médiation pénale et à la médiation familiale en cas de violences au sein du couple. Il parachève ainsi une évolution, entamée il y a plusieurs années, qui a déjà beaucoup restreint le recours à la médiation : elle ne peut à l'évidence constituer une procédure adaptée en cas de violences au sein du couple en raison de l'inégalité entre l'agresseur et sa victime. Plusieurs articles visent ensuite à alourdir les peines encourues ou à créer de nouvelles infractions. Des circonstances aggravantes sont introduites pour certains délits, quand les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS. Le délit de harcèlement du conjoint serait puni plus sévèrement lorsque le harcèlement a conduit au suicide de la victime, ce qui n'est pas rare. Il est également prévu de compléter le code pénal pour sanctionner, au titre des atteintes à la vie privée, le fait de géolocaliser un individu sans son consentement. Ces sanctions pénales seraient complétées par ce qui s'apparente à de nouvelles formes de sanctions civiles. Une disposition porte ainsi sur la décharge de l'obligation alimentaire. Elle répond à une demande forte des associations, qui veulent éviter que les enfants dont, par exemple, le père a tué la mère, soient contraints de subvenir aux besoins de leur père meurtrier. La commission en a cependant revu la rédaction, craignant qu'une décharge automatique ne pose un problème sur le plan constitutionnel, et elle a proposé que ce soit le juge pénal qui statue sur cette question dès l'étape de la condamnation. Le texte prévoit également que le juge pourra déclarer indigne de succéder celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences ou un viol sur son conjoint. Sur ce point, la commission a élargi la liste des infractions permettant de prononcer l'indignité successorale. D'autres dispositions du texte s'inscrivent davantage dans une démarche de prévention.

Certaines mesures longuement débattues au cours du Grenelle se révèlent d'une portée plus limitée. Il en est ainsi de l'article 9, sur la saisie des armes que peut posséder le conjoint violent : la saisie est déjà autorisée et pratiquée au cours des enquêtes et la proposition de loi vient seulement rendre plus lisible le cadre juridique applicable. Ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Même remarque concernant la possibilité de déroger au secret médical pour signaler des faits de violences conjugales, même en l'absence d'accord de la victime : un examen attentif montre que cette dérogation vise des hypothèses très restrictives- il faut, à la fois, un danger immédiat pour la victime et une emprise pour la victime et une emprise -, pour lesquelles il est déjà admis que le professionnel de santé puisse déroger au secret médical au nom de l'obligation de porter secours à une personne en péril. L'ajout qui nous est proposé a donc surtout un but pédagogique à destination des professionnels de santé il cherche à attirer leur attention sur la situation des femmes victimes de violences conjugales, au risque cependant de rendre plus complexes des exceptions au secret professionnel qui ne sont déjà pas toujours lisibles. J'en arrive à l'article 11 sur l'accès des mineurs aux sites pornographiques, qui a pour objet de codifier une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation et qui ne modifie donc pas l'état du droit en vigueur. vigueur. Le contrôle effectif de l'accès des mineurs à ces sites constitue pourtant un problème majeur : il n'est pas rare aujourd'hui que les mineurs aient accès à ces contenus pornographiques dès le collège, lorsque les parents leur confient leur premier smartphone.

Il avait raison ! On ne peut que s'inquiéter des conséquences que l'exposition précoce à ces images peut entraîner sur le développement psychologique et affectif de ces jeunes, et sur les relations entre garçons et filles. J'étais donc peu satisfaite du manque d'ambition de la proposition de loi sur le sujet, mais le court délai dont nous avons disposé pour l'étudier ne m'avait pas permis d'approfondir cette question avant son examen en commission. Suivant une démarche un peu inhabituelle, dont je prie mes collègues de la commission des lois de bien vouloir m'excuser, j'ai donc procédé à quelques auditions complémentaires au cours de la semaine afin de pouvoir proposer au Sénat un dispositif réellement à la hauteur des enjeux. M'inspirant d'une mesure en vigueur depuis dix ans et relative aux jeux en ligne, je vous propose de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rôle de régulation, en lui donnant le pouvoir de saisir la justice pour qu'elle ordonne le blocage de l'accès aux sites qui ne prendraient aucune mesure effective pour contrôler l'âge de ceux qui consultent leurs contenus. Je crois que seul le recours à des mesures réellement dissuasives est susceptible d'inciter les éditeurs de ces sites à agir. En proposant cet amendement, je m'inscris dans la perspective tracée par le Président de la République dans son discours devant l'Unesco du 20 novembre dernier : il avait alors donné six mois aux acteurs concernés pour trouver des solutions sur une base volontaire, sans quoi il avait estimé qu'il serait nécessaire de légiférer. Six mois plus tard, le dossier n'a pas vraiment avancé et le Gouvernement n'a pas dévoilé ses intentions. Il est donc nécessaire que la représentation nationale s'en saisisse, et c'est ce que nous allons faire. J'en termine en évoquant quelques mesures qui débordent le strict cadre de la lutte contre les violences conjugales. Nous n'avons pas été convaincus par la mesure envisagée concernant l'accès provisoire à l'aide juridictionnelle dans les procédures d'urgence, qui nous a paru présenter plus d'inconvénients que d'avantages. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de la discussion des amendements. La commission a, en revanche, approuvé les dispositions relatives au droit pour les victimes de violences de se voir remettre un certificat médical, de même que celles qui ouvrent la possibilité de prononcer certaines interdictions en complément d'une peine d'emprisonnement, ou encore la création de nouvelles infractions pour mieux sanctionner le comportement odieux qui consiste à commanditer, depuis la France, des crimes ou des délits commis commis à l'étranger afin de les visionner sur internet. En conclusion, je veux souligner que nous avons besoin, certes, de bonnes lois pour lutter efficacement contre les violences commises contre les femmes et les enfants, mais aussi d'une volonté politique implacable implacable et de moyens. Il nous faut ressentir qu'il s'agit d'une priorité absolue d'éducation et de prévention. L'État doit soutenir tous ceux- policiers, gendarmes, magistrats, éducateurs, travailleurs sociaux, -qui oeuvrent aux côtés des victimes, mais aussi aux côtés des auteurs pour aider ceux-ci à prendre conscience de leurs actes et prévenir la récidive. C'est à ce prix que nous pourrons faire vivre cet objectif qui nous rassemble et qui est au coeur de notre pacte républicain : la protection des plus fragiles.

je tiens à remercier sincèrement Mme la rapporteure ainsi que la commission des lois pour leur travail. Il y a seulement sept mois, nous débattions d'une proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. Je m'interrogeais alors sur un calendrier contestable, qui nous conduisait à débattre d'un texte alors que les conclusions du Grenelle de lutte contre les violences conjugales n'étaient pas connues. Je déplore vivement que la lutte contre les violences alimente l'inflation législative, sans permettre un véritable débat parlementaire. Cet empilement de textes disparates n'a qu'un qu'un mérite, relatif : celui de faire des violences un sujet régulier de l'agenda parlementaire, au risque, parfois, de voir sortir des décrets qui vont à l'encontre des objectifs visés. exemple celui du 27 mai dernier, synonyme de recul des droits des victimes et contre lequel les avocats spécialisés s'élèvent à juste titre. Je me félicite de ce que les dispositions de la proposition de loi mettent en oeuvre des recommandations que la délégation aux droits des femmes porte parfois depuis longtemps, notamment la nécessité absolue d'interdire toute médiation pénale en cas de violence, ou encore la remise en question de l'autorité parentale pour un conjoint violent, qui, par définition, ne peut être un bon parent. Certaines dispositions auraient pu aboutir lors de la discussion de la loi promulguée en décembre 2019. Des amendements défendus dans notre hémicycle le permettaient. Écartés au Sénat, ils ont pourtant fait partie des annonces du Gouvernement, trois semaines plus tard, lors des conclusions du Grenelle ... En matière de violences conjugales, de nombreuses avancées auraient pu être atteintes depuis longtemps, car les bonnes pratiques en la matière sont connues. Il est difficile de comprendre que, sur les 88 « homicides conjugaux » analysés par l'inspection générale de la justice dans un rapport publié en octobre 2019, une seule victime ait bénéficié d'une ordonnance de protection. Difficile d'accepter que 41 % de ces femmes aient signalé en vain au parquet et/ou aux forces de l'ordre, avant d'être tuées, des violences ou menaces qu'elles subissaient. Difficile d'admettre que 7 de ces meurtres aient été commis malgré une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Difficile, enfin, de croire que 90 % des femmes victimes de violences aient pu se déclarer satisfaites de l'accueil reçu dans les commissariats et gendarmeries, selon et gendarmeries, selon l'audit annoncé lors du Grenelle. Ce n'est absolument pas le constat fait par les experts entendus par la délégation ! La discussion de cette proposition de loi intervient après plusieurs semaines de confinement, qui ont rendu difficile la protection de femmes et d'enfants enfermés dans un foyer violent. Pendant ce confinement, notre délégation a centré son travail sur les violences. Parmi les lacunes pointées par les interlocuteurs de la délégation, citons l'insuffisante interaction entre la police, le parquet et le juge civil. Soulignons aussi la nécessité, évoquée par Luc Frémiot, ancien procureur de la République de Douai, d'encadrer plus strictement l'activité des procureurs en matière de lutte contre les violences et d'organiser, pour les auteurs de violences, un suivi psychologique dans la durée. Le principal enjeu est d'abord de permettre aux victimes que le confinement a tenues éloignées des institutions judiciaires de porter plainte. Elles ne doivent plus recevoir pour toute réponse une main courante inutile. Il est impératif de leur assurer un accueil adapté, sur tout le territoire, en métropole comme dans les outre-mer. Nous ne pouvons plus accepter que les chances d'une victime d'être crue et prise au sérieux dépendent de la sensibilisation aux violences conjugales du professionnel qui va les accueillir. la responsabilité de l'État pour faute lourde dans des affaires de violences conjugales, comme cela a été le cas à Grande-Synthe, se doit de demeurer une exception. Il y a urgence ! Pour de nombreuses femmes et de nombreux enfants, le confinement n'est pas terminé : la réalité quotidienne des familles maintenues dans une terreur permanente par un conjoint ou un père violent ressemble à un confinement sans fin. La priorité pour nous est de gagner le combat contre les violences conjugales, et de le gagner tous ensemble. Cette proposition de loi y contribuera-t-elle ? Espérons-le. Dans chaque commissariat, dans chaque gendarmerie et dans chaque juridiction, toutes les victimes de violences doivent pouvoir rencontrer des professionnels acharnés à les protéger. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons gagner ce combat ensemble ! La parole

Madame la présidente, mesdames les ministres, madame la rapporteure- je salue aussi nos collègues masculins qui participent à ces travaux, comme chaque fois que nous traitons de ce thème très important nous sommes ici réunis pour un exercice un peu particulier. Vos interventions, mesdames les ministres, l'ont bien mis en lumière. Nous débattons en

pour la troisième fois en quelques mois, un texte qui n'aura ni fait progresser les choses ni amélioré le sort des femmes et leur protection. Nous n'avons pas de retour, à ce jour, sur ce qui s'est passé pendant la période du confinement.

la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a marqué une prise de conscience à la fois sociale, judiciaire et législative de l'urgence de briser le tabou des violences conjugales, et d'y remédier par des dispositions fortes.

Un pan entier de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes aggrave les sanctions et améliore l'accompagnement des victimes à long terme : durée de l'ODP portée de quatre à six mois, maintien de la victime dans le logement du couple, meilleure protection des enfants, extension du champ d'application de l'ODP aux violences sur les enfants, possibilité de retrait total ou partiel de l'autorité parentale, restriction du recours à la médiation pénale, déploiement du téléphone d'alerte grave danger- un dispositif qui a été très utile durant le confinement, avec une forte augmentation du nombre d'attributions. Comme le disait récemment Ernestine Ronai, « lorsqu'il existe une politique publique, volontariste et claire, on obtient des résultats ». Plus récemment, nous avons examiné la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et, en novembre 2019, la loi visant à agir visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi Pradié, adoptée à l'issue du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Même si je déplore le calendrier choisi pour examiner dans l'urgence cette proposition de loi, nous devons en apprécier les nouvelles avancées. Certaines avaient déjà été proposées au vote du Sénat sous la forme d'amendements lors de l'examen de la loi Pradié. J'avais moi-même déposé des amendements en vue de restreindre l'autorité parentale ou d'empêcher le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales, conformément aux indications des juges et des pédopsychiatres auditionnés par la délégation aux droits des femmes, qui nous exhortent sans relâche à privilégier l'intérêt de l'enfant. Grâce à eux, nous savons maintenant qu'un conjoint violent ne peut pas être un bon parent. Le maintien à tout prix de l'autorité parentale, du droit de visite ou de la garde du parent violent conjugal est dénoncé unanimement, car ce sont autant d'occasions de perpétuer l'emprise sur la victime et sur l'enfant, autant de risques majeurs de sur-violence, en particulier pendant les périodes de séparation et, ajouterais-je, en période de confinement. Il n'est pas concevable qu'un parent ayant tué ou violenté son conjoint puisse continuer à exercer son autorité parentale. besoin, pour se construire, de sécurité affective et matérielle. S'il est pris dans un conflit de loyauté ou de protection, il ne peut pas le faire. Cette vérité doit franchir les portes des tribunaux et devenir une évidence judiciaire sur tout notre territoire. C'est pourquoi je salue les articles 1 et 2, satisfaits par la loi Pradié, tout comme l'article 3 suspendant le droit de visite et d'hébergement, ou encore les articles 4 et 5 interdisant la médiation pénale en cas de violences conjugales. La reconnaissance de l'emprise comme violence psychologique sera aussi un changement de paradigme déterminant pour toutes les victimes. L'article 6 décharge les enfants d'un parent condamné pour violences conjugales de l'obligation alimentaire envers celui-ci. L'article 8, autre pilier du texte, permettra aux médecins de signaler aux autorités judiciaires des violences exercées au sein du couple. C'était aussi une recommandation, martelée depuis longtemps, Avant de conclure, j'évoquerai les conséquences du récent confinement. Il nous permet de nous rendre compte que ce huis clos de violences n'est autre que la terrible réalité que vivent tous les jours, crise sanitaire ou pas, toutes les victimes de violences. Je voudrais vous citer les propos d'une victime que Luc Frémiot, ancien procureur de la République, nous a rapportés lors de son audition par la délégation aux droits des femmes, laquelle, vous le constatez, Mon mari et moi habitons au quinzième étage d'une tour. Il a calculé qu'il me fallait trois minutes pour descendre lorsque l'ascenseur fonctionne, six ou sept minutes quand je dois descendre à pied, tant de minutes pour aller au supermarché, tant de minutes pour faire ceci, tant de minutes pour revenir. Quand je suis en retard d'une minute, je suis frappée. Cela n'arrive pas qu'aux autres, et nous devons tous être des lanceurs d'alerte ! Dès le mois de mars, beaucoup a été fait pour mobiliser la population et protéger les victimes, à l'image de notre délégation qui a publié une tribune dans la presse alertant l'opinion sur l'enfer vécu par les femmes et les enfants enfermés

Des expérimentations ont été multipliées, qu'il faudra pérenniser, comme l'envoi de SMS d'alerte au 114, l'éloignement des conjoints violents du domicile conjugal vers des chambres d'hôtel, ou encore des campagnes d'affichage des numéros d'urgence. Je regrette pourtant que certains points soient absents de ce texte, tels que la lutte contre les violences incestueuses, qui sont les plus difficiles à concevoir et à nommer, jusque dans le code pénal. Or il ressort de nos auditions qu'une fille court 6,5 fois plus de risques qu'une autre personne d'être victime de violences sexuelles incestueuses si elle a un parent violent conjugal. J'avais déposé, sans succès, des amendements pour renforcer la qualification pénale des actes incestueux sur mineur. Il est urgent de briser aussi Il serait également souhaitable de prévoir une prise en charge psychologique très large des enfants témoins de violences conjugales, y compris les plus âgés et ceux qui sont issus de familles recomposées. Ils sont souvent les grands oubliés, laissés sans repères pour se reconstruire. Enfin, mes collègues du groupe RDSE et moi-même serons vigilants sur la création du nouveau comité de pilotage national annoncé par Mme la garde des sceaux pour améliorer la mise en oeuvre des ordonnances de protection. Pour autant, j'aimerais obtenir quelques explications. La collègue

aujourd'hui le tabou est bel et bien brisé. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à considérer la question de la lutte contre les violences envers les femmes comme un fil rouge de notre mandat de parlementaire. Considérant que cette proposition de loi participera à ce que la peur change de camp et contribuera à une meilleure protection des victimes de violences conjugales et de leurs enfants, mon groupe votera en faveur de ce texte. La parole

les statistiques glaçantes sur les violences conjugales viennent nous rappeler l'importance de ce fléau dans notre pays. Chaque année, en France, 220 000 femmes subissent des violences au sein de leur couple. En 2019, ce sont 150 d'entre elles qui ont perdu la vie ; elles étaient 121 en 2018 et 109 l'année d'avant. de 2017, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) rapporte que les violences intrafamiliales sont plus fréquentes et plus graves en outre-mer qu'en métropole. L'insularité et la faible superficie de certains territoires peuvent en effet entraver la libération de la parole, et rendre inopérant l'éloignement du conjoint violent ou le choix d'un lieu anonyme pour être accueillie et écoutée sans crainte. Bien sûr, je n'oublie pas que ce phénomène touche aussi les hommes, dans une moindre mesure. Fort heureusement, nous avons assisté ces derniers mois à une prise de conscience collective de l'urgence à agir contre ces faits, qui ont trop souvent été relativisés. En septembre 2019, le Gouvernement a lancé un Grenelle des violences conjugales dont la restitution des travaux, deux mois plus tard, a donné lieu à des annonces fortes. Pour tenir compte de la situation spécifique dans les outre-mer, un budget de 800 000 euros leur a été attribué. Le 28 décembre 2019, certains dispositifs annoncés, tels que la généralisation du bracelet anti-rapprochement, l'amélioration du traitement des requêtes en vue de la délivrance d'une ordonnance de protection, ou encore la suppression de l'autorité parentale, trouvaient une traduction législative lors du vote à l'unanimité de la loi Pradié. La présente proposition de loi, poursuivant ce travail, était également adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier. Au Sénat, la crise sanitaire nous a malheureusement contraints de reporter son examen, prévu initialement début avril. Pourtant, face aux circonstances inédites liées au confinement, les violences familiales ont été exacerbées et les signalements de violences conjugales ont également augmenté d'au moins 30 %, jusqu'à 36 % durant cette période. La situation étant exceptionnelle, des mesures exceptionnelles ont été mises en place par le Gouvernement pour porter secours aux victimes, mais également pour prévenir les violences : numéro d'écoute, plateforme, point d'accompagnement dans les centres commerciaux, signalement à la pharmacie, éviction du domicile du conjoint violent, Il nous revient aujourd'hui de poursuivre le travail législatif engagé par nos collègues députés. Il me semble important de souligner, à titre liminaire, que ce texte s'emploie à mieux définir dans notre droit ce que recouvre le terme de « violences », en inscrivant dans la loi la notion d'emprise psychologique, cette stratégie de contrôle qui détermine le passage à l'acte. On la retrouve à plusieurs reprises dans le texte. Ainsi, le recours à la procédure de médiation en matière civile et pénale en cas d'emprise d'un conjoint sur l'autre, ou en cas d'allégation de violences, sera écarté. De même, tout médecin ou professionnel de santé qui le souhaite pourra directement alerter le procureur de la République, sans l'accord de la victime, s'il a l'intime conviction que celle-ci est en danger immédiat et qu'elle se trouve sous l'emprise de l'auteur des violences. Cette dérogation aux règles régissant le secret médical a pu inquiéter, mais elle a été élaborée en accord avec le Conseil national de l'ordre des médecins et n'est possible que dans des conditions très restrictives. Le cybercontrôle, qui représente un moyen d'asseoir son emprise sur l'autre, est également pris en compte dans ce texte : le fait de géolocaliser une personne sans son consentement sera dorénavant sanctionné.

aujourd'hui contraindre l'ascendant ou le descendant d'une victime de crimes ou de délits commis par le créancier d'aliments. La commission des lois a considéré que l'automaticité retenue par les auteurs de ce texte présentait un risque d'inconstitutionnalité et a réécrit le dispositif. De même, il semblait important de permettre aux juges de déclarer indignes de succéder les personnes condamnées à une peine criminelle pour avoir commis des violences ou un viol envers le défunt.

Ce texte contient également des dispositions relatives à la protection des mineurs. Je pense à la possibilité accordée au juge de suspendre le droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur dans le cadre d'un contrôle judiciaire, en cas de violences conjugales, ou à la lutte contre l'exposition des mineurs à la pornographie, qui véhicule, on le sait, une image dégradée de la femme. Enfin, la proposition de loi renforce la répression de ces violences en alourdissant les peines encourues dans les cas de harcèlement sur conjoint ayant conduit au suicide, de viol du secret des correspondances téléphoniques ou encore d'usurpation d'identité du conjoint. La commission des lois a créé une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants au conjoint nous vous présenterons un amendement visant à aligner les peines encourues sur les peines graduelles qui répriment le délit de harcèlement moral du conjoint. Cette proposition de loi contient des dispositions importantes, attendues par les victimes et par la société dans son ensemble. Vous l'aurez compris, le groupe La République En Marche soutient fortement son adoption. L'engagement de la procédure accélérée démontre une volonté politique de faire reculer ces violences. Les sujets évoqués ne s'écartent pas des annonces rendues publiques par le Gouvernement, à l'issue du Grenelle, et l'urgence de la situation de ces femmes commande que nous légiférions rapidement. Évidemment, l'ensemble de ce nouvel arsenal juridique, dorénavant très complet, ne sera pleinement efficace que s'il s'accompagne d'une véritable évolution des mentalités. Nous partageons tous le même constat et nous avons les mêmes objectifs ; je ne doute pas que nous saurons trouver un point d'équilibre lors de la commission mixte paritaire

quoi de commun entre Sylvia, Bas-Rhinoise de 40 ans, Carine, 48 ans, originaire de la Loire-Atlantique et Aminata, 31 ans, résidente de la Seine-Saint-Denis ?

Sylvia est décédée après avoir demandé le divorce à son mari ; Carine a été assassinée par son ex-petit ami, qui n'avait toujours pas accepté leur rupture, intervenue pourtant deux ans auparavant Aminata, enfin, a été tuée par son conjoint et a succombé à ses blessures, sous les yeux de ses deux filles. L'urgence aurait justifié qu'un projet de loi d'envergure aborde de front

Sur le fond, nous ne sommes pas opposés à cette proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale par le groupe LaREM avec des intentions pour la Nous saluons, par exemple, les dispositions prévues aux articles 3 et 11 A, susceptibles d'accroître la sécurité des mineurs. Il en va de même de la mesure autorisant, à l'article 9, l'officier de police judiciaire à saisir, lors d'une perquisition

Ces éléments introduisent dans le XXI siècle, la lutte contre les violences faites aux femmes, ces dernières étant désormais régulièrement victimes de cyberharcèlement et de maltraitance numérique.

ce qui peut surtout être reproché à ce texte, finalement, n'est pas tant ce qu'il contient que ce qu'il omet. Nous y retrouvons les travers de la loi Pradié, promulguée en décembre 2019 : la seule réponse donnée aux violences intrafamiliales relève de la répression et le texte laisse de côté toute dimension éducative et préventive. C'est regrettable. Qu'en est-il de la formation des policiers, des magistrats et du personnel de santé ? Ces professionnels sont les premiers à recueillir les témoignages des victimes, à constater leurs blessures, à entendre leur souffrance. Ils devraient être formés

Ensuite, qu'en est-il des moyens financiers qu'il conviendrait d'allouer à cette cause ? Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 1 milliard d'euros devraient être consacrés à cette mission ; dans le projet de loi

Enfin, qu'en est-il de l'accompagnement psychologique ou, à tout le moins, de la thérapie comportementale à destination des conjoints violents ? Peut-on les guérir ? La question reste ouverte, surtout lorsqu'il s'agit, ce qui est généralement le cas, d'un comportement pervers de possession et de manipulation, qui piège la victime dans la boucle infernale de l'emprise. Accompagner les agresseurs, c'est aussi protéger les victimes. Dans un esprit constructif, le groupe CRCE déposera plusieurs amendements afin de faire évoluer cette proposition de loi. Nous tâcherons de la doter d'un volet préventif, pour équilibrer sa dimension répressive. Mes chers collègues, en dix ans, environ 1 400 femmes ont été tuées par leur compagnon leur ex-conjoint. Les femmes représentent 80 % des victimes d'homicides conjugaux ; c'est pour elles que nous légiférons aujourd'hui. Toute loi contre les violences conjugales est aussi un mémorial pour ces femmes assassinées et, plus encore, un espoir pour celles qui veulent échapper à pareille mort. Malgré nos réserves, nous voterons pour ce texte. La

dans son rapport de 2018, la délégation d'aide aux victimes a donné des chiffres d'homicides au sein du couple. Le bilan s'établit à 149 homicides, dont 121 femmes et ; à ces 149 victimes s'ajoutent 21 enfants tués dans le cadre de violences au sein du couple. Depuis lors, ces chiffres ont, bien entendu, baissé, mais ils demeurent trop importants et rappellent notre incapacité collective à protéger ces femmes, ces hommes et ces enfants, toutes ces victimes d'un conjoint, d'un ex-conjoint ou d'un parent violent, qui se transforme peu à peu en assassin. C'est pourquoi, face à cette réalité insupportable, la République doit être à la hauteur. Aussi, je me félicite de ce que le Parlement ait déjà fait évoluer la législation depuis deux ans, puisque deux textes ont été votés dans le but de combattre plus efficacement les violences commises à l'encontre des femmes et des enfants. Tout d'abord, a été adoptée la loi de 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa. Elle ne vise pas spécifiquement les violences conjugales ou intrafamiliales, mais elle contient un ensemble de mesures destinées à lutter contre les violences faites aux femmes et à mieux protéger les mineurs. Elle a notamment institué une nouvelle infraction, l'outrage sexiste, permettant de mieux sanctionner le harcèlement de rue. Elle a également élargi la définition du harcèlement en ligne. En ce qui concerne la protection des mineurs, elle a précisé la définition du viol, afin que ce crime soit plus facile à caractériser lorsque la victime est mineure, et elle a également porté le délai de prescription à trente ans à compter de la majorité de la victime. plus récente du 29 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi Pradié, porte plus spécifiquement sur les questions de violences commises au sein du couple ou au sein de la famille. Elle a donné une base légale à l'utilisation d'un nouvel outil de prévention des violences conjugales : le bracelet anti-rapprochement, dont le port peut être ordonné par le juge pénal. Ce bracelet électronique permet de prévenir la victime que son conjoint violent se rapproche et déclenche une alerte dans un centre de surveillance, afin que les forces de police ou de gendarmerie interviennent si le conjoint violent n'obtempère pas au premier avertissement. Cette loi a également renforcé le régime juridique de l'ordonnance de protection, afin que celle-ci soit délivrée dans les délais les plus brefs par le juge aux affaires familiales et que le recours au bracelet anti-rapprochement puisse être proposé dans ce cadre, de manière à prévenir la répétition des violences. La proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, qui nous est soumise cet après-midi, est donc examinée après deux lois. Ce texte fait bien sûr suite au Grenelle contre les violences conjugales, qui s'est tenu à l'automne dernier. Elle transcrit dans le droit certaines de ses préconisations, en matière civile comme pénale. Elle déborde toutefois du strict champ de la lutte contre les violences conjugales, pour inclure des mesures visant à protéger les mineurs ou à prévenir les violences au-delà du cadre des affaires intrafamiliales. Ce texte contient une série de nouvelles dispositions. Je note avec satisfaction un certain nombre de mesures, comme la suspension du droit de visite, de la médiation pénale et de la médiation familiale.

ensuite, par l'allocation de moyens aux associations qui soutiennent les victimes, enfin, par l'organisation de campagnes de communication visant à favoriser la libération de la parole.

La persistance est une meurtrissure qui ne peut être ignorée et qui nous impose d'agir. Ce combat doit mobiliser la société civile et la puissance publique. Approuvant pleinement la démarche suivie par la commission des lois, le groupe Les Indépendants votera en faveur du texte de la commission.

mesdames les ministres, mes chers collègues, 10 000, c'est le nombre d'appels qu'a reçu la plateforme 3919 durant le confinement, preuve, s'il en fallait une encore, du danger que courent les femmes dans notre société. Nous étudions aujourd'hui- cela a été dit maintes fois -le troisième texte en moins de deux ans sur les violences faites aux femmes. C'est la preuve que le temps de lutter contre ce fléau est arrivé. C'est positif, parce que cela complète utilement l'arsenal juridique dont nous disposons déjà, mais cela ne doit pas masquer le fait que cet arsenal n'est pas toujours employé, du moins suffisamment, sur notre territoire. Il est donc temps de passer de la parole aux actes. Pour autant, cette proposition de loi apporte des améliorations et elle est l'écho du Grenelle contre les violences conjugales. Certes, certains des éléments de ce texte auraient pu être adoptés dès l'examen de la proposition de loi Pradié. Certes, ce texte ne reprend pas l'ensemble des recommandations du Grenelle et il faudra sans doute un quatrième texte. Néanmoins, cette proposition de loi apporte des améliorations. On y retrouve, par exemple, la saisie des armes des conjoints violents, l'évolution du secret médical ou encore la suspension du droit de visite en cas de soupçon de violences. L'auteur du texte a également traité- c'est à saluer -des nouvelles formes de violences exercées les nouvelles technologies. Ainsi y trouve-t-on la pénalisation du cyberharcèlement entre conjoints ou encore celle de la géolocalisation non consentie. Puisque l'on parle d'informatique, je veux souligner l'évolution apportée par notre rapporteur, Marie Mercier, sur l'inscription au Fijais des individus condamnés pour consultation de contenus pornographiques. Nos travaux réalisés dans le cadre de la mission d'information sur la pédocriminalité dans les institutions avaient mis en évidence l'importance faible accordée à la consultation d'images pédopornographiques. Or cette consultation est souvent le symptôme d'un mal bien plus profond, car, ne l'oublions pas, l'enfant violé sur une image ou dans un film est un enfant véritablement violé.

Comment peut-on penser qu'il soit nécessaire et même positif de garder un lien entre le bourreau et sa victime ? Je me réjouis de constater que l'obligation alimentaire et le droit de la succession puissent être écartés en cas de crimes ou de délits intrafamiliaux. viens à la notion d'emprise ; celle-ci est maintenant reconnue. L'emprise est une mare de mazout dans laquelle on se débat. On ne peut s'en sortir seul ; il faut l'intervention d'une personne extérieure pour vous extraire du magma dans lequel vous êtes englué, pour vous aider à nettoyer vos ailes et à reprendre, ensuite, votre envol. L'emprise est souvent, malheureusement, la clé de compréhension des situations de violences répétées, qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Enfin, autre apport de ce texte : la question du secret médical et la possibilité pour un médecin d'y déroger. Naturellement, cette dérogation est encadrée et la rapporteure apporte des nuances bienvenues dans la rédaction du texte. Pour autant, à titre personnel, je défendrai un amendement sur ce sujet, car la notion retenue de « danger immédiat » pour la vie d'une victime me semble malvenue. En matière de violences conjugales, lorsqu'une victime fait face à un danger immédiat pour sa vie, il est déjà trop tard et, dans cette circonstance, on se rend rarement chez son médecin de famille ; c'est aux urgences qu'on la retrouvera, dans le meilleur des cas

la circulaire de Mme la garde des sceaux rappelant que les enfants témoins de violences conjugales sont aussi des victimes et doivent être, à ce titre, représentés ; ou encore au numéro d'appel mis en place par la Fnacav pour les hommes violents. Je me permets de rappeler, à cette occasion, que, dans le cadre de notre rapport sur la pédocriminalité dans les institutions, Marie Mercier, Michel Meunier et moi-même appelions de nos voeux un tel numéro pour les pédophiles, afin d'éviter que ceux-ci ne deviennent pédocriminels.

Une meilleure formation de ces acteurs permettrait de détecter, le plus en amont possible, ce poison. Une bonne formation des policiers et des gendarmes permettrait de mieux accueillir les victimes et de proscrire la main courante pour favoriser un dépôt de plainte systématique. maintenant évoquer les moyens, car la bonne intention n'est pas suffisante. Prenons l'exemple des stages pour les hommes violents une excellente idée sur le papier, mais, dans les faits, il y a tellement peu de places et de psychologues qu'il faut attendre plusieurs mois pour y participer, et ces stages ne durent que quelques heures, quelques jours au mieux. Pensez-vous qu'un homme qui ne communique que par la violence soit guéri en deux jours Ne croyez-vous pas que les six mois d'attente pour être traité sont six mois d'enfer pour le conjoint ? Je pourrais aussi parler du manque criant de psychologues dans les commissariats ou dans les gendarmeries, du manque d'infirmières scolaires ou encore de la baisse des aides aux associations. y a encore beaucoup de besoins à satisfaire, mais, bien sûr, ce n'est pas parce que le chemin est long qu'il ne faut pas le prendre. Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste votera ce texte.

Ce texte s'inscrit dans le prolongement du Grenelle contre les violences conjugales, ouvert par le Gouvernement le 3 septembre dernier. Il a vocation à être le complément de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, qui était issue de la proposition de loi de notre collègue député Aurélien Pradié. loi de 2019 constitue, à n'en pas douter, une véritable avancée pour les victimes, avec la possibilité donnée au juge d'ordonner la pose du bracelet anti-rapprochement, le recours élargi au téléphone grave danger ou encore le renforcement du dispositif de l'ordonnance de protection, désormais délivrée plus rapidement et plus protectrice pour les victimes. Il est, par exemple, d'une importance capitale que le conjoint violent puisse être évincé du domicile conjugal dans les plus brefs délais. Cette loi a par ailleurs prévu diverses mesures afin de faciliter le relogement des victimes de violences et il faut s'en réjouir, car le logement constitue l'élément fondateur de toute reconstruction personnelle. Alors, pourquoi ce nouveau texte est-il déposé au Parlement avant même que la loi de 2019 ait démontré la pleine mesure de sa capacité à juguler les violences conjugales et à servir durablement les victimes, sous réserve qu'elle soit assortie de financements suffisants pour soutenir les associations et les dispositifs judiciaires, comme le bracelet anti-rapprochement Permettez-moi d'y insister : la loi Pradié est un texte pragmatique, apportant des solutions juridiques précises. Ainsi, des dispositions concernant l'autorité parentale, figurant initialement dans le texte qui nous est soumis, il ne reste plus grand-chose, la commission des lois de l'Assemblée nationale a dû se résoudre à constater que la législation en vigueur traitait cette question de manière adéquate. Depuis 2014, la juridiction de jugement a en effet l'obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale de l'auteur d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de l'autre parent. Il s'agit là d'une mesure de protection de l'enfant, qui répond à la tragédie familiale qui affecte directement ce dernier. Néanmoins, les décisions de retrait de l'autorité parentale prises sur le fondement d'infractions commises sur l'autre parent étaient jusqu'ici trop peu nombreuses, sans doute parce que prévalait une certaine idée, selon laquelle l'intérêt de l'enfant réside dans le maintien, coûte que coûte, de liens familiaux avec l'auteur des violences. L'apport de la loi du 28 décembre 2019 est ici intéressant à plus d'un titre celle-ci permet désormais aux juridictions civiles et pénales, qui ont la faculté de prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, de prononcer alternativement le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, elle a prévu une suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale pour six mois, afin de libérer l'enfant de la tutelle de l'auteur du crime, dans l'attente d'une décision pérenne de l'institution judiciaire. Ces dispositions devraient rapidement faire la preuve de leur efficacité à préserver l'intégrité physique et morale des enfants, au regard d'une opinion publique tolérant de moins en moins les violences intrafamiliales et la persistance d'une certaine domination de la figure paternelle. Or ce sont justement les enfants, particulièrement vulnérables, qu'il nous faut sans relâche protéger des dérives des adultes. Notre délégation aux droits des femmes, dont je salue la vigilance constante sur tous ces sujets, a mené de nombreuses auditions sur le thème des violences intrafamiliales. Tous nos interlocuteurs ont attesté les conséquences souvent dramatiques de ces violences sur la construction identitaire des enfants. Ceux-ci sont d'autant plus fragilisés que les faits de violences sont répétés, s'aggravent et s'inscrivent dans un rapport de force asymétrique. L'impact de ces faits est variable selon le degré d'exposition à la violence conjugale, mais aussi selon l'âge et le sexe Certains experts évoquent un syndrome de stress post-traumatique pouvant être accompagné d'effets négatifs affectant le développement de l'enfant ou ses conduites : fonctionnement cognitif et émotionnel perturbé, santé dégradée, problèmes d'échec scolaire, démonstrations d'agressivité et usage de la violence. À l'âge adulte, ces enfants exposés présentent un risque bien réel de reproduire les comportements violents dont ils ont été les témoins. Toute politique publique doit donc rechercher les solutions permettant de favoriser la résilience. C'est pourquoi la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, que nous examinons aujourd'hui, me semble comporter une mesure importante au regard de cet objectif la possibilité donnée au juge de suspendre le droit de visite et d'hébergement dont une personne placée sous contrôle judiciaire est titulaire. Cette possibilité n'était pas prévue par la loi de 2019, le juge pouvant seulement prononcer à l'encontre de l'auteur des faits, dans le cadre du contrôle judiciaire, une interdiction de s'approcher de la victime et de paraître au domicile ou aux abords immédiats de celui-ci. L'exercice du droit de visite et d'hébergement est en effet un moment particulièrement redouté par les victimes de violences conjugales. Permettre au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention d'ordonner, à ce stade de la procédure pénale, la suspension du droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants est une mesure indispensable, complétant utilement le dispositif de protection des victimes. Je la soutiens donc totalement. Permettez-moi toutefois de former, au terme de cette intervention, un voeu : il est temps, me semble-t-il, de mettre un terme à cette inflation législative et de laisser l'ensemble des acteurs, en particulier ceux de la chaîne pénale, se saisir des nouveaux outils mis à leur disposition, pour combattre le fléau des violences conjugales. La parole

raillées, moquées, caricaturées dans l'histoire de notre société, mais sans qui l'on ne parlerait probablement toujours pas des violences conjugales, sans qui l'on considérerait toujours qu'il s'agit là d'une affaire privée et en aucun cas d'un sujet politique. Il faut leur rendre hommage, parce que nous n'en avons pas encore fini avec la compréhension collective du phénomène et avec l'action publique contre les violences intrafamiliales, contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

avec une coutume de la chancellerie, qui consiste à penser qu'il ne faut pas se mêler de l'office du juge. Or, plus on laisse le juge libre, en particulier en matière de justice civile et de justice familiale, plus on on multiplie les occasions que la séparation soit une occasion de violence pour les femmes. Nous présenterons des amendements tout à l'heure, qui viseront non pas à tenir la main du juge,

probablement qu'il faut laisser le juge libre. Or « le juge » n'existe pas dans la vraie vie : c'est un concept d'étudiants en droit. Dans la vraie vie, il y a des quantités de juges et des femmes maltraitées par la justice civile

le texte que nous examinons aujourd'hui est le deuxième vecteur législatif issu du Grenelle contre les violences conjugales, dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 novembre dernier. La méthode et le calendrier sont contestables, puisque nous voilà réunis pour examiner un nouveau texte quelques mois seulement après l'adoption de la proposition de loi de notre collègue de l'Assemblée nationale, Aurélien Pradié, et que nous avons eu peu de temps pour l'étudier. Cependant, il faut en souligner les avancées, malgré un arsenal juridique déjà très complet. En particulier, on peut évoquer le chapitre III, relatif aux exceptions d'indignité en cas de violences intrafamiliales, qui prévoit d'élargir le champ d'application des exceptions d'indignité en matière d'obligation alimentaire et de succession en cas de condamnation pénale. Très concrètement, l'objectif est d'éviter que des enfants dont le père aurait tué la mère ne soient légalement tenus de subvenir aux besoins de leur père au titre de l'obligation alimentaire, ce qui, sur le plan moral, nous semble, bien entendu, difficile à admettre. Cette disposition est fondamentale, puisqu'elle permet, je le crois, de renouer avec la tradition du code civil, dont l'esprit est de moraliser les comportements à travers la règle. Les précisions apportées en la matière par la commission des lois du Sénat sont bienvenues. J'y souscris. Ainsi, plutôt que de faire de la décharge de l'obligation alimentaire un automatisme, il semble plus judicieux de faire confiance à l'appréciation du juge. Il en va de même pour la possibilité désormais accordée au tribunal judiciaire de déclarer indigne de succéder une personne condamnée pour avoir commis des violences graves sur le défunt. Je salue, à cet égard, la proposition de la commission des lois d'aller plus loin sur la question, en permettant le prononcé de l'indignité successorale, quand bien même le conjoint aurait seulement été condamné à une peine correctionnelle ou serait décédé avant que l'action publique ait pu être engagée. Néanmoins, les dispositions relatives à la protection de l'enfance sont pour le moins limitées. Si la possibilité de suspendre le droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un contrôle judiciaire apparaît comme une mesure purement technique, elle vient, en réalité, combler une lacune et se révélera essentielle en pratique. En revanche, le chapitre VIII, qui porte expressément sur la protection des mineurs, contient seulement trois articles, hétérogènes et de portée limitée. À titre d'exemple, l'article 11, qui vise à protéger les mineurs contre les messages pornographiques, aura, en l'état, peu d'influence sur le droit en vigueur. Quant à l'article 11, qui incrimine le fait, pour des Français établis sur le territoire national, d'obtenir des vidéos de crimes, notamment d'abus sexuels, commis à l'étranger, il semble assez éloigné de l'objet de cette proposition de loi et met une nouvelle fois en évidence un manque de cohésion globale de la politique de protection des victimes de violences sexuelles. Notre objectif commun demeure la protection des femmes et des mineurs face aux violences perpétrées au sein de la famille. À ce stade, il semble opportun de s'interroger sur la pertinence future de l'outil législatif pour endiguer ce mal, dans la mesure où la législation française apparaît désormais comme relativement complète. Une véritable prise de conscience sociétale était nécessaire. Je veux croire qu'elle est en train de s'opérer. Personne ne doit plus jamais fermer les yeux face à une situation de violence, même si cette dernière prend place dans l'intimité du cercle familial.

Je tiens à saluer le travail considérable des associations, des professionnels du droit, du personnel médical, des partenaires privés et de tous ceux qui sont en première ligne pour concourir à la lutte contre les violences intrafamiliales et permettre ce changement profond. Je veux également saluer la délégation aux droits des femmes, qui nous permet d'auditionner régulièrement ces acteurs décisifs et de faire avancer notre réflexion et notre travail de législateur. Pour conclure, je remercie notre rapporteur, Marie Mercier, de la qualité de son travail, de son engagement et de l'humanisme dont elle a fait preuve, à chaque reprise, sur ce sujet particulièrement sensible, comme sur d'autres d'ailleurs. Lorsque l'on traite de ces questions douloureuses, nous considérons que tout texte qui concourt à une amélioration de la situation est un progrès. Je ne doute donc pas qu'un nombre significatif des membres du groupe Les Républicains, auquel j'appartiens, votera cette proposition de loi, telle qu'amendée par la commission des lois. La parole

je ne reviendrai pas sur les brutalités glaçantes et effroyables que subissent les victimes de violences conjugales. Pour les réduire, améliorer la loi a son importance. loi a son importance. Je veux à mon tour rappeler le travail qu'a déjà entrepris notre collègue Aurélien Pradié. Il a permis des avancées significatives, notamment en réduisant le délai de délivrance des ordonnances de protection et en élargissant le recours au téléphone grave danger. Je salue, bien sûr, la volonté des députés de la majorité de s'inscrire dans cette démarche, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi. Pour autant, comme beaucoup, je partage la remarque de notre rapporteur, Marie Mercier, lorsqu'elle regrette que, en l'espace de quelques mois, nous ayons eu à délibérer sur deux textes portant sur le même sujet, comme je fais mienne, après d'autres, son interrogation sur la pertinence de l'outil législatif pour endiguer un tel fléau. Appelée de longue date, la levée du secret médical pour les médecins est une avancée significative du texte. Celui-ci apportera également des progrès en matière de prévention, d'accueil, de suivi, de protection, où beaucoup reste à construire. Après la loi Pradié, il fallait que la majorité laisse sa marque législative. C'est fait- elle sera faible. Mais la loi ne réglera pas tout. Faciliter le travail des associations en l'inscrivant dans le temps, mieux former la police et la gendarmerie au repérage et à l'accueil, améliorer la réactivité de la justice, mieux coordonner l'action de tous quand il s'agit de prendre en charge la victime, de la protéger, de la loger et de l'éloigner : les enjeux Je veux, sur toutes ces problématiques, saluer les travaux de notre délégation aux droits des femmes, sous la houlette de sa présidente, Annick Billon. Depuis plusieurs mois, nous avons décidé d'aller dans nos départements, à la rencontre des associations engagées engagées auprès des victimes. Je l'ai fait dans les Pyrénées-Atlantiques. Je dois dire que j'ai découvert des hommes et des femmes solidement engagés pour apporter aux victimes soutien psychologique, juridique et matériel. J'ai découvert un dynamisme réconfortant, mais également une fragilité des structures

à des fins moins évidentes que l'assistance aux victimes. Deuxièmement, leur financement relève non pas d'un seul ministère, d'une seule direction départementale ou régionale, mais de plusieurs- justice, solidarité, intérieur, logement -, chacun avec son mode de fonctionnement, ses contraintes, son calendrier, voire ses remises en question, qui peuvent interrompre brutalement, ici, une permanence territoriale éloignée, ou, là, un accompagnement pourtant apprécié et salué. Que de temps passé en démarches ! Que d'instabilité, là où il faudrait davantage de moyens, certes, mais surtout de stabilité et de lisibilité dans la durée pour faire grandir les actions de protection en nombre et en qualité Troisièmement, ces structures sont souvent contraintes de fonctionner en silo, chacune dans leur domaine, sur leur secteur, alors que le développement de synergies serait une véritable chance pour apporter aux victimes tout le soutien nécessaire. En effet, ce type de violences est spécifique. Il exige des pouvoirs publics une protection et une prise en charge permanentes et toujours personnalisées. Le nombre de décès pour cause de violences conjugales qui surviennent alors que la victime s'était signalée nous oblige à rechercher une perpétuelle amélioration. Celle-ci passe non pas uniquement par la loi, mais par des moyens mieux coordonnés et des procédures simplifiées. À ce titre, les collectivités territoriales, par leur proximité, devraient, à mon sens, jouer un rôle plus important. J'en forme le voeu. Pour autant, malgré sa faiblesse et parce qu'elle est dans le prolongement de la proposition de loi, issue de notre famille politique, entrée en vigueur à l'hiver dernier, le groupe Les Républicains

déjà à l'oeuvre avec beaucoup de volontarisme. Je veux simplement évoquer un point qu'a soulevé Mme de la Gontrie, à propos du décret publié le 28 mai dernier, dont l'objet était d'assurer la mise en oeuvre des ordonnances de protection

Notre objectif premier- vous le savez, madame de la Gontrie -est bien entendu de multiplier la délivrance des ordonnances de protection, parce que nous considérons que cet outil juridique peut être extrêmement protecteur pour les femmes.

Je veux être très claire avec vous : dès demain, la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes de mon ministère réunira des professionnels. Elle réunira également les associations concernées. En outre, comme je l'ai dit, je mets en place un comité de pilotage, de suivi des ordonnances de protection. Je n'aurai aucune difficulté à prendre en compte les suggestions qui pourraient m'être formulées et les rectifications qui apparaîtraient nécessaires. Bien évidemment, si celles-ci semblent judicieuses et respectent le principe du contradictoire, je rectifierai le texte rapidement et sans hésitation. Mon seul souci est l'effectivité de la délivrance des ordonnances de protection.

La lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales nécessite des moyens à la hauteur des ambitions affichées. Les dispositions de la présente proposition de loi ne seront efficaces que si que si le Gouvernement renforce de manière importante les moyens de la justice et des associations intervenant dans le domaine des violences conjugales. Les moyens et les modalités d'intervention de la police et de la formation de l'ensemble des professionnels de la justice, de la police, des services sociaux, médicaux et de l'hébergement devront être évalués. Par ailleurs, cette lutte ne sera efficace qu'avec une information massive sur les outils mis à la disposition des victimes. L'objet du présent amendement est donc d'assurer une bonne information des parlementaires sur les moyens consacrés par le Gouvernement aux politiques de lutte contre les violences conjugales. Quel est l'avis de la commission ? la commission est, par principe, réservée sur les demandes de rapport. En l'espèce, il semble que beaucoup d'informations sont déjà disponibles, le sujet des violences conjugales ayant été largement débattu ces derniers mois. Par ailleurs, il s'agit d'un sujet dont le Parlement pourrait se saisir, par exemple, par le biais de la délégation aux droits des femmes, ce qui serait plus profitable que de demander au Gouvernement d'évaluer sa propre politique. Au-delà de cette demande de rapport, je sais que notre collègue souhaite, par ce biais, évoquer la question des moyens, qui n'est pas facile à aborder directement compte tenu de l'application de l'article 40 de la Constitution. Il s'agit bien sûr d'une question majeure : l'accueil des victimes, la prise en charge des auteurs, le soutien au milieu associatif, les solutions d'hébergement sont des priorités qui nécessitent des moyens à la hauteur. Par conséquent, la commission est défavorable à l'amendement lui-même, mais reconnaît une convergence de vues sur le message que nos collègues souhaitent faire passer à l'occasion de ce débat.

que « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale ». L'adoption de cet amendement n'est donc pas utile et pourrait même créer un risque d'interprétation, en donnant l'impression que, pour d'autres infractions, une main courante pourrait se substituer au dépôt de plainte, ce qui serait contre-productif.

de nombreuses femmes sont venues nous expliquer que, lorsqu'elles ont voulu déposer plainte, on leur a proposé de faire une main courante. Ignorant le code de procédure pénale, les malheureuses ont cru,

Si nous éprouvons le besoin de le répéter, c'est parce que nous sommes désarmés devant la résistance d'un certain nombre de services de police ou de gendarmerie, qui continuent de penser que la main courante est suffisante en cas de violences conjugales.

le déclenchement d'une enquête et le signalement auprès du parquet. Il me semble que, psychologiquement, il peut être utile que les victimes aient à leur disposition

pour explication de vote. Nous partageons l'argumentaire de Mme de la Gontrie : il est indéniable que les nouvelles règles de fonctionnement fixées par le décret du 27 mai 2020 en ce qui concerne l'obtention d'une ordonnance de protection représentent un danger pour les victimes de violences conjugales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, madame la garde des sceaux, nous proposions également, dans notre amendement n° 84, jugé irrecevable en vertu de l'article 41 de la Constitution, que l'ordonnance soit notifiée au défendeur par le ministère public- que ce dernier soit ou non à l'initiative de la requête. Nous sommes tout à fait conscients de la difficulté de légiférer en la matière. Il s'agissait tout de même de rectifier la procédure de notification de l'ordonnance de protection

L'administration nous a fait savoir qu'une proposition de réécriture avait été proposée à nos collègues socialistes. Nous nous en réjouissons, mais nous n'avons pu bénéficier de la même faveur, car notre amendement reprenait des alinéas du décret. J'entends le sujet, mais, hélas, ce n'est pas la première fois que l'application des irrecevabilités ne joue pas en notre faveur. À un moment, mes chers collègues, il faudra refaire le point sur cette pratique pour faire en sorte qu'elle s'applique dans les mêmes termes, quel que soit le groupe à l'initiative des propositions d'amendements.

question a trait au partage des compétences entre le Gouvernement et le législateur : il ne s'agit en aucun cas d'une appréciation sur les mérites de votre amendement.

en intégrant clairement les violences psychologiques, définies à l'article 222-14-3 du code pénal, à l'ordonnance de protection. Le caractère psychologique des violences- menaces, dévalorisation de l'autre, insultes, rabaissement récurrent, isolement ... -participe de l'installation du phénomène d'emprise de l'auteur des violences sur la victime.

Or les associations spécialisées et les avocats amenés à accompagner les femmes victimes de violences commises par leur conjoint ou ancien conjoint soulignent tous un manque de prise en considération du caractère psychologique des violences. Cet amendement a donc pour objet de renforcer la prise en charge de tous les mécanismes de la violence conjugale.

de la vraisemblance de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés d'interprétation. En effet, cette rédaction sous-entend que le danger n'est pas forcément produit par la violence, et donc qu'il y aurait des violences sans danger. Cela pousse certains praticiens à écarter l'octroi de l'ordonnance de protection en considérant que les violences alléguées ne constituent pas un danger suffisant. Cette situation engendre un risque pour de nombreuses femmes. Toute violence doit entraîner une protection de la victime. Le présent amendement vise donc à rendre plus effective la portée de l'ordonnance de protection en supprimant cette exigence cumulative.

est à Mme Monique Lubin. Pour la délivrance des ordonnances de protection, la notion de « danger » est souvent interprétée par les juges du fond comme un danger de moins de huit jours auquel est exposée la victime. Or le danger qui peut se déduire des faits de violences allégués peut s'analyser en danger vraisemblable et non en danger actuel caractérisé. Le danger doit être présumé avec la vraisemblance des violences. Cet amendement, proposé par le

de repli par rapport au précédent, remonte des professionnels, en particulier des professions judiciaires qui accompagnent les femmes victimes de violences. Il est fondé sur la pratique.

? Cet amendement tend à prévoir que le JAF statue obligatoirement sur chacune des mesures qu'il peut prononcer dans le cadre de l'ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties.

En pratique, il n'est appliqué qu'à titre subsidiaire, et est trop peu sollicité. Le présent amendement vise à améliorer l'effectivité de ce principe, les victimes n'ayant plus à faire la demande de leur maintien dans le logement. Sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, le maintien au domicile de la personne qui n'est pas l'auteur des violences est de droit.

Il me semble que nous étions arrivés, à l'époque, à un équilibre satisfaisant en inscrivant clairement dans la loi que le logement du couple est attribué à la personne qui n'est pas l'auteur des violences et que, si le juge souhaite déroger à ce principe- vous vous en souvenez -, il doit satisfaire à une double exigence en justifiant de circonstances particulières et en motivant spécialement sa décision. Priver le juge de tout pouvoir d'appréciation

Le présent amendement est inspiré des recommandations des associations d'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Partant du principe qu'un conjoint violent n'est pas un bon père, ses auteurs souhaitent prévoir l'examen systématique,

de l'autorité parentale de la partie défenderesse, puis sur les modalités du droit de visite et d'hébergement. La suspension de l'autorité parentale n'entraîne toutefois pas automatiquement la cessation de la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, ni celle de l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un PACS, de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, comme le prévoit actuellement l'article 515-11 ; d'où les modifications prévues par le présent amendement au 5° dudit article, en cohérence avec le dispositif prévu au 1° de

Le JAF peut- je le rappelle -se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce qui permet de protéger l'enfant et le conjoint victime. Lui confier un pouvoir de suspension de l'autorité parentale dans le cadre de l'ordonnance de protection ne nous semble pas opportun. Nous avons voté, il y a à peine quelques mois, un autre mécanisme, de suspension

être très attentif : je me permets d'être précise -, pour six mois, pour les personnes poursuivies ou condamnées, même non définitivement, pour un crime sur l'autre parent. Je rappelle qu'en outre les parents violents peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale,

qui a fait l'objet d'une mesure d'éviction du domicile et d'une mesure d'éloignement, mais qui conserve le droit, parce qu'il a et exerce l'autorité parentale, de savoir où ses enfants sont scolarisés,

de lever l'anonymat du domicile de la mère et des enfants. C'est pourquoi nous proposons que, dans l'ordonnance de protection, le juge puisse aussi prévoir que le lieu de scolarisation des enfants n'est pas communiqué au père qui, pour autant, a conservé l'exercice de l'autorité parentale. de l'autorité parentale. Quel est l'avis de la commission ? Comme vous l'avez bien précisé, ma chère collègue, le présent amendement tend à permettre au JAF d'autoriser la victime de violences à dissimuler l'adresse de l'établissement scolaire des enfants dans le cadre d'une ordonnance de protection. Il s'agit là de retirer à l'un des parents l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale. Mais les deux sont liés : si et seulement si le juge confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des deux parents, alors il est possible de priver l'autre de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. S'il n'a plus

bien entendu, l'adresse de l'école ne figure pas et ne doit pas figurer dans l'ordonnance de protection. Mais si vous visez une dissimulation du nom de l'établissement scolaire en dehors de toute procédure, celle-ci se rattache en réalité à la question de l'exercice de l'autorité parentale

si le juge a organisé l'exercice de l'autorité parentale de telle façon que le père violent n'exerce pas cette autorité pendant la durée de l'ordonnance de protection, on peut effectivement imaginer que, dans ce cas-là, ce dernier n'ait pas connaissance de l'adresse des enfants. Mais la justice, en France, est très réticente

le père a le droit- c'est un droit -de savoir où sont scolarisés ses enfants. S'il téléphone à la mairie ou au rectorat, il peut le savoir. Autrement dit, on exfiltre une femme et ses enfants, on dissimule son adresse, mais on conserve au père le droit de savoir où les enfants sont scolarisés et, ainsi, on lui conserve ouvert le chemin pour arriver jusqu'à la mère.

L'ordonnance de protection ne présente pas les mêmes garanties qu'un jugement : on va vite parce qu'on croit qu'il y a un danger ; on est convaincu qu'il vaut mieux prendre le risque de se tromper en protégeant cette femme contre un danger que de prendre le risque de ne pas la protéger. Mais quand on en arrive à des mesures plus complètes, alors il faut respecter le contradictoire. Il ne suffit pas d'alléguer des violences pour déclencher des décisions de manière systématique, sans respect des droits de la défense. Faites attention, je vous en conjure : à vouloir multiplier les réglages textuels de pure procédure, vous n'améliorerez en rien la protection des femmes ! Quand le juge veut prendre des mesures protectrices, il a à sa disposition tout un arsenal de mesures à prendre. En l'occurrence, pour ne pas donner l'adresse de l'école des enfants, il a déjà tout ce qu'il faut. de vote. Je veux simplement dire au président Bas que ce n'est pas parce que c'est une ordonnance qu'il n'y a pas de contradictoire. d'ailleurs parlé longuement : c'est justement pour ce motif de respect du contradictoire que le délai de six jours est si compliqué à respecter. J'indique d'ailleurs qu'il est possible de faire appel. Nous ne sommes pas d'accord : certains pensent que, pour protéger une femme, une mère, il faut, dans certaines circonstances que seul le juge peut apprécier, que le lieu de scolarisation de l'enfant ne soit pas connu du père violent ; d'autres ne le pensent pas. Mais ne cherchons pas des arguties procédurales

Lorsque la victime de violences obtient le bénéfice d'une ordonnance de protection, le conjoint ou ex-conjoint auteur des violences peut être exclu du logement à ce titre. Or, actuellement, dans l'hypothèse où l'auteur des violences est titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire, et ce de manière unilatérale, la résiliation ou la rupture du contrat de bail. Cette situation n'est que trop fréquente. Cet amendement vise à s'assurer, d'une part, que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail, et, d'autre part, que le bailleur ne puisse le rompre qu'avec l'accord exprès de la victime qui occupe le logement. Ainsi, l'ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime.

Votre amendement pose plusieurs difficultés. Le dispositif proposé fait mention du logement commun ou conjugal. Or les époux sont automatiquement cotitulaires du bail ; dans cette hypothèse, aucune résiliation unilatérale du bail n'est possible.

: celui-ci n'a pas connaissance des décisions judiciaires et, surtout, il n'a aucune relation contractuelle avec la personne qui n'est pas titulaire du bail- il ne la connaît même pas. En tout état de cause, une personne victime de violences à laquelle le JAF attribuerait la jouissance du logement ne pourrait pas être expulsée de ce logement, une telle mesure ne pouvant être prononcée telle mesure ne pouvant être prononcée que par un juge. La victime bénéficiaire d'une ordonnance de protection ne serait pas considérée comme sans droit ni titre, et il n'est pas imaginable qu'un juge prononce l'expulsion dans ce cas-là. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

en faveur de l'attribution des logements en urgence aux personnes qui sont victimes de violences. Ce n'est pas le sujet que vous évoquez, madame la sénatrice, mais c'est tout de même un point important dans la gestion de ces questions de logement. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

à la présence des enfants et de prévoir que l'ordonnance de protection sera toujours communiquée au procureur de la République. Quel est l'avis de la commission ? ? Le présent amendement tend à systématiser l'information du procureur de la République de toutes les ordonnances de protection qui sont délivrées. Le parquet est en principe tenu informé, car il est présent à tous les stades de l'instance civile. Il reçoit toutes les demandes d'ordonnance de protection et il est partie jointe à l'audience dans la plupart des cas. La loi ne prévoit toutefois son information expresse lors de la délivrance d'une ordonnance de protection que dans le cas particulier d'enfants en danger. Compte tenu des difficultés qui ont pu être relevées dans les circuits d'information entre magistrats il me semble qu'effectivement il pourrait être utile de préciser dans la loi que toutes les ordonnances de protection font l'objet d'une information sans délai du parquet. Je ne crois pas qu'une telle mesure affaiblisse la protection des enfants. La commission émet donc un avis favorable.

votre amendement produirait l'effet contraire de l'objectif visé. Ah ! Aussi, je voudrais vous convaincre de le retirer. Comme vous le savez, toutes les décisions en matière d'ordonnance de protection, qu'elles acceptent ou qu'elles rejettent la demande, sont déjà communiquées au procureur de la République,

C'est le parquet qui fait procéder à l'inscription de l'ordonnance de protection au fichier des personnes recherchées et au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes si la décision est prise en ce sens. Il en a donc nécessairement connaissance. Vous souhaitiez que le parquet soit toujours informé, mais, je vous le réaffirme ici, c'est déjà le cas. votre amendement tend à supprimer l'information spécifique du procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger. La disposition que vous voulez abroger prévoit en effet un signalement spécial concernant les mineurs en danger

mais je n'ai absolument rien entendu qui permette de limiter le champ d'information du parquet. Je souhaite donc vraiment que cet amendement soit adopté : ainsi, les parquetiers seront toujours informés des ordonnances de protection.

réserve la transmission de l'ordonnance de protection au parquet à la seule hypothèse où il y aurait des parents violents susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. C'est bien ainsi que nous interprétons tous l'article 515-11 du code civil, madame la garde des sceaux sur ce point à cet instant, madame la garde des sceaux ? L'article 515-11 du code civil prévoit aujourd'hui que la transmission au parquet de l'ordonnance de protection est réservée à l'hypothèse dans laquelle il y aurait des violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants

sceaux. Je ne veux pas avoir l'air de m'opposer pour m'opposer, mais je dis simplement que, depuis la loi Pradié, il est précisé à l'article 515-10 que le ministère public est informé systématiquement de toutes les ordonnances de protection. Nous avons expressément souhaité laisser dans l'article 515-11 un signalement quand il y a un enfant en danger, parce que c'est une alerte supplémentaire, un signalement tout particulier

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre mois à six mois ce délai. Les mesures de l'ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée, ou si le juge a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale pour la durée de la procédure. Je considère qu'il s'agit d'un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l'atteinte aux libertés individuelles. L'ordonnance de protection est un outil de l'urgence, dont il faut renforcer l'efficacité, mais cela ne peut pas, si les violences persistent et que des infractions sont commises, remplacer une procédure pénale,

mois à six mois en 2014. Surtout, comme vous le savez, l'ordonnance de protection est prolongée de manière automatique et systématique, sans nouvelle décision du juge, dès lors qu'il y a une demande en divorce, en séparation de corps ou sur l'exercice de l'autorité parentale. Il me semble que ces

: La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi. Afin de mieux protéger les victimes, la loi du 28 décembre 2019 a utilement permis au juge aux affaires familiales de prononcer le port du bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l'ordonnance de protection. Pour autant, l'article 511-11-1 du code civil, tel qu'il est issu de cette loi, rattache le prononcé du bracelet anti-rapprochement à l'interdiction de contact avec la victime, sans toutefois le lier à une interdiction de s'en approcher, qui fragilise la portée du dispositif. En effet, les forces de l'ordre ne peuvent dès lors intervenir qu'une fois que les interdictions de contact ou de paraître ont été effectivement violées. Le temps d'intervention des forces de l'ordre en est retardé, et la protection de la victime, par là même, éprouvée. Il s'agit là d'un point non négligeable, qui doit appeler notre vigilance, mes chers collègues. C'est pourquoi nous proposons de mentionner, au sein du code civil, que le JAF qui ordonne le port d'un bracelet anti-rapprochement aura, au préalable, interdit à l'auteur des violences de s'approcher à moins d'une certaine distance de la victime. Cette modification permettrait d'assurer une assise légale à l'intervention des forces de l'ordre lorsque le porteur d'un bracelet anti-rapprochement se maintient dans la zone après le déclenchement d'une première alerte. En conclusion, il s'agit d'assurer la pleine efficacité du dispositif que notre assemblée a adopté à la fin de l'année dernière, avec l'objectif, que nous partageons tous ici, de la protection effective des victimes.

au ministère qui travaillent sur le bracelet anti-rapprochement, puisque cela fait partie des engagements forts que mon ministère avait pris, et qui ont été ensuite inscrits dans le cadre de la loi du 28 décembre dernier. Nous venons, au moment où je vous parle, d'envoyer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) le décret qui va permettre la mise en oeuvre de ce bracelet anti-rapprochement. C'est une étape qui est absolument nécessaire, puisque, évidemment, le traitement de ce dispositif suppose un fichier informatisé, qui doit donc recevoir l'avis de la CNIL.

meilleurs et des plus performants lieux d'expertise sur les mécanismes des violences faites aux femmes et sur les féminicides. La FNSF nous demande de prévoir que le parent bénéficiaire d'une ordonnance de protection ne soit pas tenu de communiquer à l'autre parent tout changement de résidence lorsqu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il s'agit encore de renforcer la protection du parent victime pendant la période de l'ordonnance de protection, en lui évitant de devoir informer l'autre parent

l'avis de la commission ? Cet amendement est similaire à l'amendement n° 71, que nous avons examiné tout à l'heure à propos de la dissimulation du lieu de scolarisation des enfants. C'est la même problématique : il s'agit de retirer à l'un des parents l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale, à savoir connaître le lieu de résidence de son enfant. Il n'est donc possible de le faire que si le juge retire l'exercice de l'autorité parentale au défendeur dans l'ordonnance de protection. Si le juge confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des deux parents,

pour la commission de faits de violence sur l'autre parent ou sur l'un des enfants ? Aujourd'hui, c'est possible ! On vous dira : « liberté du juge », « appréciation du magistrat », « pouvoir d'appréciation des circonstances

parent. Quel est l'avis de la commission ? Là encore, nous devons faire preuve de réalisme. Cet amendement vise à interdire au juge de fixer la résidence principale d'un enfant chez un parent condamné pour des faits de violences à l'encontre de l'autre parent ou de ses enfants. Par principe, la commission souhaite laisser au JAF le soin d'apprécier chaque situation et de décider dans chaque cas, en fonction de l'intérêt de l'enfant. C'est cela, juger ! Les pratiques des JAF évoluent. Les nombreux travaux récents les ont sensibilisés sur l'impact des violences conjugales sur les enfants et remettent en cause l'idée qu'il faudrait à tout prix distinguer le mari violent du père. Par ailleurs, l'interdiction proposée ne semble pas proportionnée, car elle vise tout type de condamnation et n'est pas limitée dans le temps. Je vais vous donner un exemple : une condamnation est prononcée lorsque l'enfant a 2 ans en l'état de la rédaction de l'amendement, cette interdiction serait maintenue, par exemple, jusqu'à ce qu'il devienne un adolescent de 15 ans. La loi du 29 décembre 2019 a déjà créé de nouveaux dispositifs qui permettent au juge de suspendre l'exercice de l'autorité parentale au moment d'une condamnation pour crime ou délit, ou même de suspendre de manière automatique l'exercice de l'autorité parentale pour les crimes dès les poursuites ou la condamnation. Une telle suspension empêche que la résidence principale soit fixée chez le parent condamné ou poursuivi.

les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. À partir de là, il me semble que le juge fera le meilleur choix possible sur la fixation de la résidence ou l'autorité parentale.

tout à fait dommageable pour la justice, mais aussi pour les enfants, que nous imposions une décision automatiquement, alors qu'elle doit être pesée

la rigueur de la loi, en créant un automatisme, empêche le juge aux affaires familiales de prendre la mesure qui, dans ces cas, et uniquement

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

par la délégation aux droits des femmes le 20 mai dernier, à savoir que la mère victime de violences conjugales se voit attribuer exclusivement l'exercice de l'autorité parentale.

Une interdiction qui serait totale et absolue de l'exercice des droits parentaux par effet de la loi, sans contrôle effectif qui puisse être fait ni de la proportionnalité par les tribunaux du type d'infraction commise ni de l'intérêt des mineurs, ne serait pas, me semble-t-il,

des parents qui ne respectent pas le jugement de séparation ou le jugement sur l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque le

c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Évidemment, si Mme la garde des sceaux me dit qu'elle est favorable à cet amendement, je le

Les débats que nous venons d'avoir le démontrent. Une remise à plat de l'ensemble des dispositions du code civil sur l'autorité parentale serait souhaitable. Celles-ci restent marquées par le principe de coparentalité et ne permettent pas, en dépit des avancées législatives récentes, de tirer les conséquences des violences conjugales.

pourquoi subordonner la suspension de plein droit de l'autorité parentale pour le conjoint violent à la commission d'un crime contre l'autre parent ? Pourquoi ne pas remettre en cause son autorité, du fait même qu'il exerce des violences contre son conjoint ? Les spécialistes le savent : le premier besoin des enfants est la sécurité et la stabilité, ainsi que l'a indiqué à la délégation un magistrat auditionné pendant le confinement. Il faut inscrire dans le code civil l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale en cas de violences conjugales au parent victime. Il faut également que le code civil évolue, pour que l'auteur de violences conjugales ne puisse rencontrer son enfant que dans un espace de rencontre et en présence d'un tiers. Il est nécessaire d'adopter des règles simples fondées sur des principes simples. Cette proposition de loi est donc une avancée, mais une avancée incomplète. C'est pourquoi cet amendement vise à faire en sorte que la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ne soient pas limités à une période de six mois.

présumées innocentes tant que le jugement n'a pas été donné. L'amendement n° 79 vise à limiter la suspension de l'exercice de l'autorité parentale jusqu'au procès en cour d'assises.

Nous pensons qu'il est raisonnable de laisser vivre cette loi avant de l'amender.

que le juge exprime une motivation spéciale, lorsqu'il décide de maintenir le droit de visite et d'hébergement, malgré les violences exercées auparavant par le père sur la mère des enfants.

sans qu'il y ait besoin de rechercher l'intention de l'auteur des faits, pour que la sanction soit prononcée. Enfin, c'est un délit pour lequel le demandeur peut utiliser la citation directe.

de son affaire. Quel est l'avis de la commission ? La citation directe est une procédure qui permet à la victime de surmonter une éventuelle inertie

est à Mme Annick Billon. La législation actuelle suspend l'application des obligations liées à la mise à l'épreuve pendant le temps de la détention. Dès lors, les interdictions de contact qui ont pu être imposées par la juridiction de jugement n'entrent en vigueur qu'à la libération du condamné. Cette suspension peut mettre en danger la victime, dans la mesure où le chef d'établissement pénitentiaire a la liberté d'accorder un parloir ou une unité de vie familiale pendant le temps de détention du condamné, risquant de maintenir le phénomène d'emprise. On sait que de nombreux conjoints continuent depuis leur cellule à terroriser leur compagne et, à travers elle, leurs enfants. La détention peut donc n'offrir aux victimes aucun répit. Il est nécessaire de mettre fin à cette incohérence difficilement compréhensible. Les contacts entre le conjoint violent et sa victime peuvent être interdits quand l'auteur de violences n'est pas incarcéré, mais ils sont possibles pendant la détention. Quel est l'avis de la commission ? Il semble

d'ailleurs déjà évoqué ce sujet devant vous et précisé qu'un décret modifiant l'article D. 403 du code de procédure pénale était en cours d'écriture. Il est est destiné à prévoir une telle interdiction : chaque fois qu'une interdiction de contact aura été décidée par une juridiction, quel qu'en soit le cadre, elle empêchera la délivrance d'un permis de visite.

En revanche, supprimer le délit de non-représentation d'enfant me semble excessif. Dans un certain nombre de cas, nous l'avons bien vu, la non-représentation d'enfant est extrêmement douloureuse

donc indispensable de conserver ce délit, autrement dit cette pénalisation d'un comportement inacceptable. Je vous rappelle par ailleurs que, juridiquement, on ne peut pas poursuivre du chef de non-représentation d'enfant la personne qui agirait en état de nécessité. La jurisprudence admet que, lorsqu'il existe un danger actuel ou imminent pour l'enfant, la personne qui ne le remet pas ne sera pas pénalement responsable du délit de non-représentation d'enfant. En outre, si l'intérêt En outre, si l'intérêt de l'enfant est de ne pas voir l'un ou l'autre de ses parents, il appartient au juge aux affaires familiales, dans le cadre des compétences dont il dispose,

portent sur l'étape cruciale de la libération, ou encore à l'article 745 sur le sursis avec mise à l'épreuve. D'une manière générale, il découle du caractère contradictoire de la procédure une information de la victime à différentes étapes.

Le comportement parfois déroutant de la victime ne peut en effet se comprendre que par cette notion, qui nécessite un vrai « décodage ». Comme l'a expliqué la psychiatre Marie-France Hirigoyen du Sénat : l'emprise est « une manipulation qui s'installe dans la durée, qui va conduire une femme à perdre son esprit critique ». Après l'étape de séduction, qui vise à ôter à la femme toute résistance, surviennent les propos méprisants et dévalorisants, destinés à casser la confiance en soi de la victime. Parallèlement, celle-ci subit un isolement croissant. Elle quitte son travail, ne voit plus ses amis ni sa famille, et sa vie sociale disparaît. Elle n'a plus personne vers qui se tourner. Le contrôle est également très important dans l'emprise. Il est d'ailleurs rendu plus facile par les nouvelles technologies. Ces étapes successives de l'emprise conduisent la femme à considérer que ce qu'elle vit est normal. Et, comme le soulignait le docteur Hirigoyen, la femme régulièrement battue en vient à relativiser, à nier. La médiation est, par le fait, tronquée sous l'emprise d'un conjoint violent. Cet article, qui prévoit d'exclure toute mesure de médiation en cas d'emprise, marque donc une nouvelle étape par rapport à la loi de décembre 2019, qui avait interdit la médiation dans le contexte de violences alléguées, y compris dans l'hypothèse d'une acceptation de la médiation par les conjoints, conformément à une demande ancienne de la délégation. Nous nous réjouissons donc de cet article.

N'interdire la médiation que dans les cas où elle serait manifeste apparaît trop restrictif au regard de la réalité du phénomène vécue par les victimes. De plus, laisser un champ plus large à sa définition permettra de mieux protéger les victimes dans le cadre d'une procédure civile. Ainsi- je suis sûr que les membres de la commission des lois apprécieront -, le juge pourra librement apprécier l'existence de l'emprise, sans être tenu par son caractère manifeste. Enfin, la notion d'emprise apparaissant pour la première fois dans une loi, il ne semble pas nécessaire de lui adjoindre d'ores et déjà un qualificatif restreignant son champ d'application. Pour l'ensemble de ces raisons, et par cohérence avec nos précédents

Loin de produire l'effet escompté, cette mesure nourrit plutôt une fausse impression d'impunité chez l'agresseur, qui ne mesure alors nullement la gravité de ses actes. Pour les victimes, le sentiment d'insécurité se fait plus fort, et nombre d'entre elles font ensuite l'objet de représailles de la part du compagnon contre qui elles ont porté plainte. Il semble donc qu'un simple rappel à la loi soit purement et simplement inefficace, ni répressif ni éducatif. Il ouvre plutôt la voie à une récidive des actes violents et met de ce fait la victime en danger. Le présent amendement vise à qu'un rappel à la loi pour violences conjugales soit systématiquement accompagné d'une formation de prévention et de lutte contre les brutalités au sein du couple ou d'un stage de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Si le profil de l'agresseur s'y prête, devrait également lui être proposée, afin de soigner des attitudes colériques et pathologiques. Ces mesures viseraient à responsabiliser l'agresseur,

des conjoints violents qui avaient accompli un stage perlé sur plusieurs semaines et qui témoignaient de ce qu'il leur avait apporté. Je vous réponds par un exemple, et je sais bien qu'un exemple ne vaut pas généralité, mais je puis vous assurer que c'est évidemment par des stages de responsabilisation et des thérapies que nous pouvons avancer dans la prise en charge des conjoints violents. Vous me dites, madame la sénatrice Cohen, qu'il faudrait que la loi soit plus précise. Je ne pense pas que la durée de tels stages relève de la loi.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe de travail « Justice » du Grenelle des violences conjugales l'a particulièrement mis en lumière, la décharge de l'obligation alimentaire sécurise et protège les débiteurs en cas de violences conjugales. il s'agit non pas d'interdire aux débiteurs de mettre en oeuvre cette obligation, mais d'empêcher qu'un juge ne lui ordonne de le faire. Nous proposons, avec cet amendement, de réintroduire l'automaticité de la décharge en cas de crime sur un débiteur ou sur ses proches. Toutefois, il s'agit non pas d'un rétablissement sec de l'article adopté par l'Assemblée nationale, mais d'une rédaction de compromis, sur un sujet dont nous comprenons les enjeux et la complexité. Ainsi, la rédaction que nous proposons que nous proposons ménage, comme en matière de retrait de l'autorité parentale ou de placement de l'enfant, la faculté pour le juge de prendre une décision contraire. Ensuite, elle écarte le risque d'inconstitutionnalité en ne visant que les condamnations pour crimes, respectant la hiérarchie des infractions. Enfin, conformément à la volonté de notre rapporteur, elle étant la décharge de l'obligation à l'ensemble des débiteurs d'aliments touchés par un drame familial, ce qui constitue un apport bienvenu. Nous pensons que cette rédaction offre un certain équilibre garantissant la proportionnalité du dispositif, tout en évitant que n'interviennent des situations tristement ubuesques. l'avis de la commission ? L'amendement n° 85 de Thani Mohamed Soilihi tend à rétablir le caractère automatique de la dispense de l'obligation alimentaire en cas de condamnation du créancier pour crime sur le débiteur ou ses proches, tout en prévoyant la possibilité pour le juge aux affaires familiales, saisi le cas échéant des années après par le créancier, de revenir sur cette peine automatique. je ne suis pas convaincue par votre dispositif, pour deux raisons. Malgré une atténuation, la décharge de l'obligation alimentaire reste automatique à raison d'une condamnation pénale criminelle et pose toujours un problème de constitutionnalité. Certes, vous permettez au JAF d'en relever le condamné si celui-ci le saisit d'une action en réclamation d'aliments, mais ce dispositif ne garantit pas l'appréciation ou l'intervention du juge dans un délai raisonnable. Réserver cette automaticité aux crimes ne la rend pas plus conforme à la Constitution.

interprétation du juge, une sorte de présomption en faveur du créancier, selon laquelle les délits ne constitueraient pas un manquement suffisamment grave pour justifier une décharge de l'obligation. Et comme le législateur n'élargit pas non plus la liste des « proches » du débiteur, le juge pourrait en conclure que la disposition se veut d'interprétation stricte.

je souscris à l'ensemble des motifs de votre exposé. Je pense comme vous qu'une décharge automatique, systématique et définitive de la dette alimentaire en cas de crime comme de délit sans intervention du juge serait disproportionnée. En outre, comme votre commission des lois l'a rappelé, une telle disposition, au regard de son étendue et de son caractère systématique, serait fragile sur le plan constitutionnel. Mais la rédaction de votre amendement permet précisément de mieux protéger les débiteurs d'aliments dans les cas les plus graves, les crimes, tout en conservant au juge son pouvoir d'appréciation dans le temps ou en cas de changement de circonstances, ce qui est également conforme à la volonté de la commission des lois, à laquelle j'attache la plus grande importance.

pouvoir d'appréciation. Rien ne justifierait que ce ne soit pas le cas ici aussi. De plus, la rédaction que vous proposez prend en compte l'ensemble des crimes commis sur les ascendants, descendants, frères et soeurs des débiteurs. Cet élargissement correspond à notre volonté commune de prendre en compte toutes les violences familiales. À cet égard, le texte adopté par votre commission, qui confie au juge pénal le soin de prononcer la dispense de l'obligation alimentaire, m'apparaît plus restrictif. Il permet bien sûr au juge de dispenser les débiteurs de leurs obligations alimentaires en cas de violence, mais le juge ne pourra le faire qu'à l'égard des débiteurs qui sont parties à l'instance pénale. Bien souvent, ce n'est pas le cas des enfants dans les procès pour violences conjugales ou pour viol entre époux. Dans ces cas, les enfants ne pourraient donc pas bénéficier de cette décharge. Monsieur le sénateur, votre rédaction nous permet de couvrir l'ensemble des situations. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis favorable

Mme le rapporteur. Il s'agit d'une précision rédactionnelle, afin d'exclure les condamnations pour violences volontaires de nature contraventionnelle. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mohamed Soilihi. Notre commission des lois a étendu à plusieurs cas de condamnation pour délit la faculté du juge de déclarer une indignité successorale. Je salue à ce titre l'amendement de Mme la rapporteure, qui a finalement exclu du champ des causes d'indignité les condamnations pour violences volontaires, constitutives d'une contravention. Notre amendement tend à s'inscrire dans la continuité de celui de la rapporteure, tout en allant un peu plus loin dans la logique, et sans pour autant rétablir la rédaction de l'article, telle qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale. En effet, il vise à réduire au cas de condamnation pour crime envers le défunt n'ayant pas entraîné sa mort la faculté du juge de déclarer une indignité successorale. Cette rédaction nous semble comporter au moins deux avantages. Bien qu'elle soit limitée aux crimes, elle permet de couvrir de nombreux actes graves tels que les violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, qui sont punies d'une peine criminelle lorsqu'elles sont commises par le conjoint. Par ailleurs, en étant justement limitée aux crimes, cette rédaction permet d'encadrer strictement le champ d'appréciation du juge et limite le risque de créer un nouveau champ de contentieux entre héritiers successoraux.

car, dans certaines circonstances, ces délits peuvent être suffisamment graves pour justifier une indignité. Par ailleurs, la commission a ajouté ce cas d'indignité parmi ceux qui peuvent être prononcés lorsque l'action publique a pris fin avant qu'une condamnation ne soit prononcée du fait du décès du prévenu. L'avis de

simplement répondre à Mme la rapporteure Marie Mercier, puisque j'ai manqué de courtoisie en ne le faisant pas, mais les deux sont liés. Je rappelle simplement que l'Assemblée nationale a souhaité introduire un nouveau cas d'indignité successorale facultative qui permette au juge de déclarer indigne de succéder l'héritier ayant été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol envers le défunt. Vous aviez souhaité, madame la rapporteure, élargir cette liste en y ajoutant les violences volontaires de nature correctionnelle, en excluant toutefois celles qui sont de nature contraventionnelle. Malgré cette précision, le résultat de votre amendement me semblait trop large, puisque les violences contraventionnelles peuvent devenir des délits, du fait de la circonstance aggravante de faits commis sur le conjoint. Je suis donc plutôt favorable à l'amendement de M. Mohamed Soilihi, qui tend à limiter la liste des infractions aux peines criminelles et me semble être une rédaction de compromis entre la disposition de l'Assemblée nationale et ce qui vient d'être ici proposé.

Les règles successorales entraînent souvent des non-sens lorsqu'une personne est tuée par son conjoint. En effet, présumé innocent, le conjoint de la personne décédée est souvent l'héritier direct, alors même qu'il peut être celui à l'origine du décès. Les familles sont alors doublement touchées : par la perte de leur parent et par le fait de voir l'assassin percevoir une éventuelle assurance vie ou un héritage. Dans la législation actuelle, il est prévu une exclusion automatique de la succession en cas de meurtre ou de violences ayant entraîné la mort, mais rien n'est fait en amont, et rien n'est prévu durant une enquête en cours. Le présent amendement a donc pour objet que les notaires et les organismes d'assurance vie puissent être informés des enquêtes en cours pour homicide sur conjoint. En pareil cas, le règlement de la succession ou l'application du contrat d'assurance vie doit être suspendu.

Contrairement à ce que son objet indique, le dispositif proposé ne règle pas la question en amont de l'information des notaires et des organismes d'assurance vie des enquêtes en cours, qui est la condition nécessaire pour suspendre la succession ou le règlement de l'assurance vie, vie, sur laquelle des points d'amélioration pourraient sans doute être trouvés. Dans la pratique, un notaire est informé des circonstances de la mort de la personne dont il ouvre la succession et il peut en informer à son tour l'organisme d'assurance vie. J'émets donc un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

puisqu'il vise à ajouter aux dispositions actuelles la possibilité pour la personne bénéficiaire de dissimuler son adresse, ainsi que celle de l'école de ses enfants. Bien entendu, il est cohérent avec d'autres amendements que nous avons défendus précédemment.

Quel est l'avis de la commission ? soit si l'auteur des violences a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l'ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF. De plus, si l'ordonnance de protection n'est pas en place, le procureur a déjà la possibilité de la demander, ce qui permet au JAF de se prononcer sur l'autorité parentale. Le JAF peut déjà à tout moment, pendant la durée de l'ordonnance, statuer à nouveau sur l'exercice de l'autorité parentale et sur toutes les mesures de l'ordonnance à la demande du parquet ou de l'une des parties. L'avis de la commission est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

parole est à Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences conjugales particulièrement menacées d'obtenir une identité d'emprunt. Ce dispositif, par ailleurs prévu dans le cadre de la protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions, est particulièrement lourd dans sa mise en oeuvre. Il emporte de graves conséquences dans la vie de la personne qui se saisit de cette possibilité, mais pour laquelle la disparition est nécessaire pour sauver sa vie. Actuellement, l'identité d'emprunt n'est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Notre objectif est donc de prévoir, pour les femmes en situation de grave danger du fait de leur conjoint ou ex- conjoint violent, un statut de protection supplémentaire, matérialisé par une identité d'emprunt qui leur permettrait de se dissimuler plus efficacement. La situation de menace est parfois instaurée par l'entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l'ordonnance de protection.

Ces personnes peuvent en effet craindre des représailles de la part de criminels agissant en bande organisée. Il est vrai que certaines victimes de violences conjugales peuvent craindre d'être victimes de représailles de la part de leur conjoint, notamment au moment du dépôt de plainte. Il nous semble cependant que d'autres dispositifs, comme le bracelet anti-rapprochement, peuvent leur offrir une protection plus appropriée

sauf lorsque les époux sont séparés de corps et autorisés à résider séparément, ne peut donner lieu à des poursuites pénales. Une seule exception existe jusqu'à présent, à savoir le vol portant sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité ou des moyens de paiement.

ce champ, afin que les entraves à la liberté de se déplacer, comme le vol de clés de voiture par l'un des conjoints au préjudice de la victime de violences conjugales, puissent également faire l'objet de poursuites pénales.

commis entre conjoints ou entre descendants et ascendants. Cette immunité familiale ne s'applique cependant pas aux objets ou documents indispensables à la vie quotidienne des victimes. Mon cher collègue, il semble

Meunier. Madame la ministre, et seulement les époux, car le code civil dispose que chacun d'eux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. S'il est aisé de démontrer que l'usage d'un papier d'identité par un conjoint qui n'en est pas titulaire peut avoir un caractère frauduleux, il est en revanche plus délicat de soutenir qu'un conjoint qui se comporterait comme le maître et le possesseur d'un véhicule appartenant à la communauté commettrait un vol. Cette notion de liberté de déplacement, qui pourrait recouvrir une longue liste d'objets susceptibles d'appartenir à la communauté, trouverait donc très difficilement à s'appliquer. Il me semble que les contestations que vous évoquez trouvent leur solution naturelle auprès du juge civil lors de la séparation des époux. Par ailleurs, la rédaction de cet amendement aboutirait au contraire de l'objectif puisqu'elle réprime non pas le vol des objets nécessaires au déplacement de la personne, mais le vol des objets qui entraveraient la liberté de déplacement. Pour ces différentes raisons, j'émets un avis défavorable. Monsieur Brisson,

est à Mme Claudine Lepage. Les victimes de violences conjugales peuvent souhaiter quitter le logement familial le plus rapidement possible, afin d'échapper aux coups de leur agresseur. Cet amendement a pour objet de les y aider en prévoyant pour les victimes locataires une nouvelle possibilité de réduction du délai de préavis à un mois au lieu de trois. Une telle réduction du délai de préavis est déjà prévue pour pallier certaines vulnérabilités financières liées à la santé ou encore à l'emploi. nous sommes tous d'accord, dans cet hémicycle, pour considérer que les victimes de violences intrafamiliales sont en situation de vulnérabilité. Il me semblerait logique d'accorder à tout locataire victime de telles violences un délai de préavis réduit, afin qu'il puisse quitter son logement au plus vite.

d'un délai de préavis de congé réduit sur la base d'un dépôt de plainte ou de la délivrance d'une ordonnance de protection. Il est évidemment tout à fait bien intentionné, et j'en comprends la logique, mais il existe déjà des mesures qui permettent aux victimes de violences conjugales de quitter le logement. Par exemple, lorsqu'elles doivent quitter le logement en raison des violences exercées au sein du couple ou sur les enfants, la loi portant évolution du logement, est venue renforcer leur protection en mettant fin à la clause de solidarité entre les cotitulaires du bail. La question du préavis, dès lors, ne se pose plus. Les victimes bénéficient également des cas prévus dans la loi de 1989 pour un délai de préavis réduit, notamment lorsqu'elles quittent leur logement pour un logement social. Par ailleurs, le dépôt d'une plainte n'est pas une décision de justice permettant de sécuriser le fait générateur d'une telle mesure dérogatoire au droit commun. Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.

L'hébergement des victimes de violences conjugales est une problématique constante. La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre ouvrant la possibilité à des organismes déclarés de louer des habitations à loyer modéré, afin de les sous-louer aux victimes de violences conjugales. Toutefois, le dispositif est réservé aux décisions prises dans le cadre d'un divorce ou d'une ordonnance de protection.

C'est pourquoi le présent amendement vise à étendre cette possibilité d'hébergement des victimes de violences conjugales aux concubins en intégrant au dispositif les procédures de séparation.

au sein de la famille a créé deux expérimentations relatives au logement d'une durée de trois ans. La première permet la sous-location à titre temporaire de logements du parc locatif social. La seconde ouvre un dispositif d'aide personnalisée d'accès au logement.

Cet amendement vise à élargir les expérimentations aux personnes en cours de procédure pénale ou de séparation. Or une expérimentation a pour objet de pouvoir tester un nouveau mécanisme auprès d'une population bien définie,